La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 2 octobre 2024 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n’y a pas d’observation

que l’université des sciences et technologies de Gaziantep, qui vient de rendre un hommage vibrant à Ismaïl Haniyeh, l’ancien chef du Hamas, avec 250 000 euros en prime

vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie le mercredi 2 octobre 2024, sont consultables sur le site du Sénat.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

En effet, la situation de nos finances publiques détermine nos marges de manœuvre face aux multiples défis de notre époque, qu’ils soient économiques, sociaux, démographiques, environnementaux ou géopolitiques. L’actualité nous le démontre. c’est de notre trajectoire budgétaire que dépend notre crédibilité lors des discussions avec nos partenaires européens. Or, alors même que l’immense majorité des États membres ont consenti d’importants efforts de redressement dans la période récente, la Commission européenne nous a placés en procédure de déficit excessif. Nous sommes devenus le mauvais élève. En tant que rapporteur spécial de la commission des finances pour les crédits de la mission « Engagements financiers de l’État », j’ai pu mesurer les conséquences très concrètes de notre endettement public sur le budget de la

Pour être tout à fait exact, il a progressé de 360 milliards d’euros sous la présidence de François Hollande et de 120 milliards d’euros durant les deux premières années de la présidence d’Emmanuel Macron.

Voilà la réalité. Eh ben… Rapporté au PIB, notre ratio de dette, de 112 % au deuxième trimestre de 2024, affiche certes une légère baisse par rapport au pic observé en 2021. Toutefois, son maintien à un niveau élevé, pour ne pas dire sa remontée récente, singularise fortement notre pays, que – je le répète – les autres États de la zone euro ont repris des trajectoires de désendettement très rigoureuses. Je pense en particulier à plusieurs pays d’Europe du Sud, qui se trouvaient dans des situations très difficiles et qui ont fait les efforts nécessaires.

des dépenses du ministère de l’éducation nationale, notre premier poste budgétaire. À terme, si cette trajectoire haussière n’est pas maîtrisée, les intérêts de la dette pourraient absorber en totalité le produit de l’impôt sur le revenu.

C’est un effort exigeant, dont l’ampleur est à la mesure de la situation. Vous l’avez dit : notre pays a accumulé une dette qui s’élève désormais à 3 200 milliards d’euros, représentant 112 % de notre PIB au deuxième trimestre de 2024.

: derrière ces chiffres, il y a à la fois un enjeu de soutenabilité et un enjeu de souveraineté. Il y a un enjeu de soutenabilité, d’abord, parce que la donne a changé. L’alourdissement de la charge de la dette s’explique moins par l’augmentation de l’endettement que par la forte hausse des taux d’intérêt.

Ne nous y trompons pas : cette évolution résulte également d’une dégradation de la signature France. En témoigne le nouveau creusement de l’écart de taux d’emprunt entre l’Allemagne et la France : cet écart est passé de 0,5 % au début de l’année 2024 à environ 0,8 % aujourd’hui.

Face à ces crises, nous avons choisi, de manière résolument transpartisane, de déployer un filet de sécurité parmi les plus efficaces et les plus généreux d’Europe.

il est tout aussi vrai d’affirmer que le PIB a progressé de 569 milliards d’euros sur la même période. À titre de comparaison, le taux d’endettement de notre pays a progressé de trente quatre points de PIB entre 2007 et 2017, contre seulement douze points de PIB entre 2017 et 2022.

demain. En outre, si nous ne reconstituons pas aujourd’hui nos marges de manœuvre budgétaires, comment pourrons nous, demain, protéger notre pays face à de nouvelles crises, par exemple face à une autre pandémie

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France se retrouvera t elle au bord du gouffre ? C’est la question que pose le Premier ministre et que nous pouvons légitimement nous poser. De dérapage en dérapage, l’illusion d’une bonne tenue des comptes publics s’est dissipée. Pis, la gestion calamiteuse de nos finances publiques, doublée d’un mensonge, est avérée.

Résultat : la France affiche un des déficits les plus élevés de la zone euro. La dette publique atteint 3 228 milliards d’euros, soit plus de 112 % du PIB. Quant au service de la dette, il dépasse désormais 50 milliards d’euros, devenant notre deuxième poste budgétaire.

tel constat révèle l’échec d’une politique de l’offre menée tambour battant depuis sept ans. Cette politique est fondée sur la croyance que des baisses d’impôt couplées à des aides massives aux entreprises favorisent l’emploi et la croissance.

sont, pour beaucoup, des emplois peu qualifiés, qui ont induit de faibles recettes fiscales. Pendant cette période, la productivité de la France s’est même dégradée de six points. un décrochage de la productivité, c’est un décrochage de la croissance et des recettes fiscales. Le Conseil d’analyse économique (CAE) estimait en 2019 que cette baisse de productivité représentait 140 milliards d’euros de PIB et 65 milliards d’euros de pertes Les conséquences de cette gestion calamiteuse n’ont pas tardé : la Commission européenne a ouvert une procédure pour déficit excessif contre la France. La crédibilité de la signature française est affectée et notre capacité à investir pour répondre aux urgences climatiques et sociales se réduit. Chaque euro dédié au service de la dette est un euro de moins pour nos services publics.

vous supprimerez des dépenses utiles pour nos concitoyens, celles qui soutiennent leur consommation et la croissance. Le Trésor précise d’ailleurs qu’une baisse de 15

est sujette à caution : plusieurs rapports ont mis en lumière leur manque de ciblage et leur coût exorbitant pour la puissance publique. Les élus du groupe SER feront des propositions pour rompre avec le dogme des baisses d’impôt et renouer avec la justice fiscale. Là est bien l’erreur originelle de la politique conduite depuis sept ans. Monsieur le ministre, une question demeure : après avoir accumulé des milliards d’euros de dettes, sacrifié nos services publics et compromis les investissements dans la transition écologique, comment pouvez vous encore affirmer que votre politique

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour un débat constructif sur un sujet si important que celui de l’état des finances publiques de la Nation, encore faudrait il s’accorder sur les chiffres de départ. Lorsque nous devions voter le budget pour 2024, l’hiver dernier, le Gouvernement nous promettait un niveau de déficit public à 4,5 % du PIB et un effort de maîtrise « à l’euro près » des dépenses publiques. Et puis, au cours du premier semestre de 2024, Bercy a purement et simplement annulé 10 milliards d’euros de crédits et des rumeurs de dérapage du déficit à plus de 5 % se sont fait entendre. À l’époque, déjà, Bercy refusait de transmettre au Parlement les documents budgétaires nécessaires au légitime contrôle de l’action du Gouvernement. Et puis, le 26 juillet dernier, l’Union européenne a lancé une procédure pour déficit public excessif contre notre pays. Et puis, dans son discours de politique générale, le Premier ministre nous annonce qu’en réalité, le déficit public est supérieur à 6 %, pour un montant de dette record à 3 228 milliards d’euros – pour l’instant. En définitive, le bilan du Mozart de la finance, c’est une France qui emprunte sur les marchés à des taux supérieurs à ceux de la Grèce, en faillite il y a encore dix ans, c’est 400 milliards de prestations sociales additionnelles, c’est 1 000 milliards de dette supplémentaires alors que nos services publics sont malmenés. Ces chiffres sont implacables.

Enfin, ce n’est ni aux retraités ni aux ménages français de payer votre incompétence. Faites des économies sur ceux qui profitent des largesses de notre système : je parle, par exemple, du coût de l’immigration, ou encore de la fraude fiscale et sociale – nous demandons depuis longtemps, au Rassemblement national, notamment la mise en place de la carte Vitale biométrique.

Le Gouvernement cherche des pistes d’économies ? En voici une, de taille : il est temps de mettre fin à cette folie qui consiste à engraisser avec l’impôt des Français des associations dont l’objectif avoué est d’empêcher la reconduite à la frontière des clandestins Quand j’entends le ministre du budget nous dire fièrement, à cette tribune, que l’augmentation de la dette de 1 000 milliards d’euros résulte de choix politiques pertinents et bons, les bras m’en tombent. Quand je l’entends parler de souveraineté alors que cette dette est largement détenue par des fonds souverains étrangers, je m’étouffe. Quand j’entends le ministre du budget s’exprimer, digne représentant de la Macronie, je me dis que, décidément, le nouveau monde n’a toujours pas entendu le cri de colère d’un peuple français qui l’a pourtant largement désavoué, à trois reprises, il y a à peine plus de quatre mois. L’alternance, vite ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux vous parler d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps là, en France, la dette publique avoisine les 60 % du PIB et le déficit est maîtrisé autour des 3 %. Outre Rhin, la situation est à peu près la même. En ce début du XXI siècle, la France et l’Allemagne respectent chacune les critères de Maastricht. C’est le moins que l’on puisse attendre du couple franco allemand : qu’il donne l’exemple au niveau européen. Aujourd’hui, notre dette publique dépasse les 100 % du PIB et le déficit public s’est durablement installé au dessus de 5 %. Le Gouvernement présentera jeudi le projet de loi de finances pour 2025. L’effort pour réduire le déficit est annoncé entre 45 et 60 milliards d’euros, selon que l’on compare avec le budget exécuté cette année ou avec un budget qui n’a jamais existé et qui, je l’espère, n’existera jamais… Quelle que soit l’année de référence, l’effort, monsieur le ministre, doit reposer bien davantage sur les dépenses que sur les recettes.

Si nous en sommes arrivés là, c’est que, pendant plus d’un demi siècle, la France a voté des budgets en déficit. Cette incurie est une faute collective, faut maintenant corriger. La solution la plus évidente serait de voter un budget à l’équilibre, voire en excédent. Mais ce remède, un brin radical, j’en conviens, risquerait en fait d’être pire que le mal. Car Car le mal profond, mes chers collègues, c’est l’addiction chronique à la dépense publique. Et après cinquante ans d’accoutumance, on se soigne non du jour au lendemain, mais de façon progressive. Suivons la devise des médecins : « D’abord, ne pas nuire. Le chemin sera long et douloureux – il est de notre responsabilité de le dire. Nous sommes nombreux, au Sénat, à tenir ce langage, et ce depuis plusieurs années. Je pense, bien sûr, à notre rapporteur général, Jean François Husson, qui a toujours fait preuve de constance en la matière, ainsi qu’à son prédécesseur, qui vient de s’exprimer. Pour ne pas dévier de ce cap, pour tenir bon, nous devons dire et répéter une vérité : la croissance de la dette menace notre souveraineté. Notre dette est détenue à plus de 50 % par des acteurs étrangers.

le plus sûr, en la matière, c’est qu’un créancier, qu’il soit français ou étranger, tient d’abord et surtout à être payé. Or c’est notre devoir que de payer nos dettes. Mais là réside l’ineptie de la situation : chaque titre émis par le Trésor est une obligation faite aux contribuables français de payer des créanciers étrangers, qui n’est pas la meilleure façon d’employer les deniers publics… La charge de la dette sera bientôt le premier budget de l’État, comme M. le ministre l’a esquissé. Nous consacrerons alors plus d’argent à rembourser nos créanciers qu’à payer nos enseignants, nos médecins et nos militaires. Cette situation, intenable, prépare le terrain à des solutions plus radicales et, sans doute, moins souhaitables. Pour les éviter, il faut, de toute urgence, bifurquer vers la décroissance.

C’est le seul chemin qui nous éloigne de la crise. Il est à notre portée. La preuve, c’est que nous l’avons pris, sous le gouvernement d’Édouard Philippe, de 2017 à 2019. La France sortait de la procédure pour déficit excessif en ramenant son déficit sous la barre des 3 % du PIB. La dette était stabilisée

dont seule une partie résulte des crises que le pays a traversées. De ce point de vue, la France fait clairement partie des mauvais élèves européens. Regardons la réalité en face : en 2017, la France était le sixième pays le plus endetté de la zone euro alors qu’aujourd’hui, seules la Grèce et l’Italie sont devant nous.

la trajectoire budgétaire sur de bons rails. Dans ces circonstances, s’endetter pour investir est particulièrement efficace à court terme, en maintenant la croissance, et à long terme, pour renforcer le potentiel de l’économie.

Cette question est indissociable de celle de la crédibilité de notre trajectoire budgétaire. Les économistes qui s’étaient penchés sur la question des seuils critiques de dette publique à partir desquels la croissance du PIB et la

respecter la trajectoire que l’on s’est fixée constitue inévitablement un grave et important signal d’alarme pour les marchés. Or c’est exactement ce qui s’est passé dans notre pays. Du fait de la mauvaise gestion budgétaire de la France, la dette est devenue un sérieux problème.

un niveau de déficit de 3 % du PIB en 2027, dégradent nos conditions d’emprunt. Il nous faut donc emprunter plus et dans de moins bonnes conditions, ce qui ne fera qu’accroître la charge de la dette.

Ainsi, en septembre, le taux à dix ans de la France rejoignait celui de l’Espagne, tandis que les taux à cinq ans du Portugal et de la Grèce, deux pays qui

préconisait d’« éviter des hausses de programme de financement trop importantes pour pouvoir être absorbées par la base d’investisseurs sans dégradation des conditions de financement », précisant que « cette dernière contrainte risqu[ait] d’être plus forte que la contrainte européenne

serait il pas opportun de recourir à une part de financement hors marché, compte tenu notamment du niveau d’épargne des Français ? La France a déjà eu recours

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dire la vérité exige de reconnaître les faits tels qu’ils sont. Reconnaître que, pour la fin du deuxième trimestre de l’année 2024, la dette publique de la France s’établit à plus de 3 228 milliards d’euros selon l’Insee. Dire également que, ces sept dernières années, le taux d’endettement français a progressivement augmenté, pour atteindre 112 % du produit intérieur brut en 2024, contre 98,1 % en 2017. Alors oui, l’état dans lequel se trouvent nos comptes publics doit nous préoccuper et faire comme si de rien n’était serait tout simplement irresponsable. Mais dire la vérité, toute la vérité, exige aussi de contextualiser et d’expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à une telle situation. Il est exact d’affirmer que le taux d’endettement français progresse, mais il faut revenir en arrière, bien avant 2017, pour en trouver le point de départ. En réalité, selon les données d’Eurostat et de Fipeco, la dette publique française, en pourcentage du PIB, n’a cessé d’augmenter depuis 2007. Certes, il y a eu des périodes de stabilisation, entre 1997 et 2007 et de 2016 à 2019. Mais si l’on met de côté ces moments où la dette a pu être maîtrisée, force est de constater que celle ci n’a pas connu de diminution importante depuis les années 1980. S’agissant de la dette publique brute, nous sommes ainsi passés de 21,1 % du PIB en 1980 à 110,7 % du PIB à la fin du premier trimestre de l’année 2024. Cela ne vous a pas échappé, mes chers collègues : la dette de la France a dépassé les 100 % du PIB pour la troisième année consécutive. Mais dans quel contexte ? Celui d’une période où notre pays a dû affronter les conséquences économiques de la pandémie de covid 19, de la guerre en Ukraine et de l’inflation, trois crises majeures, différentes à bien des égards, mais qui ont eu pour point commun de créer des difficultés considérables pour notre économie, tant pour nos entreprises que pour nos concitoyens. Alors oui, face aux risques catastrophiques qui existaient, les gouvernements successifs, sous l’impulsion du Président de la République, ont privilégié la sauvegarde et la protection de milliers d’entreprises, le maintien du salaire de millions de Français, avec une contrepartie inévitable : celle de l’endettement. Très bien ! Mes chers collègues, dire la vérité, c’est aussi se demander dans quel état serait notre économie si nous n’avions pas fait ces choix. Fallait il moins s’endetter, au risque de voir le chômage augmenter, les faillites se multiplier et les factures d’énergie flamber davantage, comme ce fut le cas chez bon nombre de nos voisins européens ? Certes, nous devons reconnaître que tout n’a pas été parfait. Il fallait faire vite et certaines mesures ont été prises dans l’urgence. Cependant, je suis fier d’avoir soutenu des gouvernements qui ont eu le courage de prendre des décisions difficiles, mais responsables. Reconnaissez aussi, mes chers collègues, que cet hémicycle a bien souvent soutenu les décisions budgétaires liées à la politique du « quoi qu’il en coûte », qui était nécessaire. À l’époque, parmi vous, qui a dit que nous dépensions trop ? trop ? J’entendais même parfois que nous n’en faisions pas assez. Cette crise étant désormais passée, nous devons maintenant relever le défi immense de la réduction de notre dette actuelle, un défi nécessaire, inévitable et, surtout, collectif. collectif. Je constate que la notion de « responsabilité budgétaire » semble faire consensus dans nos prises de parole. J’espère donc qu’elle se traduira concrètement dans nos actes et dans nos votes, à plus forte raison lors de l’examen du projet de loi de finances à venir.

? Bravo ! Nous n’avons pas à rougir de notre bilan. Le plan de relance et le fonds vert étaient nécessaires, et je suis fier de les avoir soutenus. S’il est un sujet que je défends, c’est la politique de l’offre menée depuis sept ans. Nous avons fait baisser le chômage, qui n’est plus un sujet, ou presque.

! En ce cas, j’ose espérer que je n’entendrai plus dire, lors des questions d’actualité au Gouvernement ou de l’examen des missions budgétaires, que le compte n’y est pas et que l’on ne crée pas assez d’emplois dans la santé, la sécurité ou la justice. Le groupe La Poste a, par exemple, annoncé une coupe budgétaire de 50 millions d’euros dans le contrat de présence territoriale qui le lie à l’État, lequel finance ses 17 000 antennes en France.

que devra désormais réaliser l’État face à l’impératif de réduction de la dépense publique. Ainsi, comment réduire les dépenses publiques tout en améliorant la qualité de nos services publics ? Autrement dit, comment dépenser moins, mais aussi, et surtout, comment dépenser mieux ? Nos concitoyens sont inquiets, exigeants, et ils veulent savoir, à juste titre, où vont et à quoi servent leurs impôts. propos en commission, monsieur le rapporteur général, puisque la situation l’exige et que les Français attendent de nous de la responsabilité, j’espère, mes chers collègues, que nous pourrons aborder collectivement l’examen du budget avec une volonté constructive et un esprit d’ouverture. Ainsi pourrons nous voter ensemble des propositions d’économies et des mesures de justice fiscale indispensables à la réduction de notre dette publique.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la dette publique et le déficit sont de véritables marronniers parlementaires, de vieux marronniers, même, puisque voilà cinquante ans que nous n’équilibrons pas nos comptes publics. Nous collectionnons, en la matière, les médailles d’or aux jeux Olympiques de la finance. Cocorico !

Dans sa déclaration de politique générale, le nouveau Premier ministre s’est engagé à ramener le déficit de la France à 3 % en… 2029. Or, en 2007, le Premier ministre d’alors, M. Fillon, parlait d’un État en faillite

qui « les dettes d’aujourd’hui sont les impôts de demain ». En la matière, les réveils sont douloureux, alors mieux vaut ne pas s’endormir…

exercices imposés pour les parlementaires que nous sommes, ne sont que rarement, voire jamais respectées, parce que les prévisions macroéconomiques sont de plus en plus aléatoires au gré des crises sanitaires ou de la géopolitique mondiale, mais surtout – surtout

Pour la France et pour nos enfants, nous devons y croire. Alors je me réfère au conseil amical de Blaise Pascal,

Le déficit annihile la liberté », dit notre ami l’inoxydable Jean Arthuis. Le réveil est difficile, mais prévisible, après des années de taux négatifs et leur effet totalement anesthésiant, comme l’a rappelé le rapporteur de la mission « Engagements financiers de l’État

ailleurs, comment comptez vous gérer les engagements hors bilan, qui représentaient plus de 3 756 milliards d’euros au 31 décembre 2023 ? Le moment est aussi venu de rappeler les positions fortes de notre groupe. Nous étions opposés à la suppression de la

également depuis plusieurs années l’encadrement des prix de transfert et bien d’autres mesures pour lutter contre la fraude sociale, dont certaines, victoire de l’optimisme sur l’expérience, sont entrées dans notre droit positif.

je ne crois pas du tout qu’il faille aujourd’hui procéder à cette opération. Pour conclure, mes collègues Michel Canévet, Sylvie Vermeillet, Vincent Capo Canellas, Vincent Delahaye, Jean Marie Mizzon,

Bocquet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il était une fois le grand méchant loup de la dette publique. Les discours anxiogènes redoublent d’intensité dans la période récente et la préparation du budget 2025 est très tendue. À l’évidence, les gouvernements successifs cherchent non pas à faire réfléchir la population, mais à lui faire peur. Le dernier budget équilibré de notre pays date de cinquante ans exactement : c’était en 1974. années plus tard, le pouvoir s’est donné un budget financé pour une moitié par les impôts et les taxes, pour l’autre moitié par de la dette. Cette année, l’État va emprunter 285 milliards d’euros sur les marchés financiers : un record historique. 150 milliards d’euros serviront à équilibrer le budget et 135 milliards à rembourser les emprunts arrivés à terme. J’ai parfois l’impression que la République française est cliente chez Sofinco, Cetelem ou Cofidis. Dans le même temps, nous paierons à nos créanciers la jolie somme de 55 milliards d’euros d’intérêts ce monde marche sur la tête – ou sur la dette ! Nos gouvernants nous expliquent que nous dépensons trop, que nous vivons au dessus de nos moyens. Pour notre part, nous avons regardé du côté des recettes

Certes, on nous explique que la TVA compensera les pertes. Toutefois, la TVA représentait 47,3 % des recettes de l’État en 2017 ; aujourd’hui, ce chiffre a chuté à 27 %. Le déséquilibre, le déficit est donc davantage dû à un problème de recettes manquantes, selon nous. Le discours anxiogène s’accompagne aussi de propos culpabilisateurs. Nous serions l’horrible génération de profiteurs… C’est vrai ! … qui s’endettent sur le dos de leurs enfants et petits enfants. Quelle honte ! Et pourtant, c’est bien nous qui remboursons la dette

% : c’était le résultat non pas d’une politique de réduction de la dépense publique, mais, bien au contraire, d’une politique de croissance et d’investissements tant publics que privés. Dans ces années d’après guerre, vouées à la reconstruction, c’est la Banque de France, avec son réseau de banques partenaires, qui formait le circuit du Trésor. Celui ci collectait l’épargne des Français et faisait des avances à l’État. C’était un système vertueux qui nous protégeait de l’emprise des marchés financiers. Or il fut démantelé progressivement au tournant des années 1970 et 1980. Mes chers collègues, connaissez vous le montant total de notre épargne ? Selon la Banque de France, les placements financiers de la Nation représentent aujourd’hui 6 111 milliards d’euros. N’y aurait il pas là une piste à explorer pour inventer un autre système de financement de l’État ? Le rapporteur général lui même y a fait référence lors de son intervention. Enfin, je

Elle détient aujourd’hui 25 % de la dette française. Autrement dit, la BCE s’est affranchie de ses propres règles, parce qu’il y avait le feu dans la maison économique mondiale. N’est ce pas le moment de poser le débat sur un rôle nouveau que pourrait jouer la BCE dans le financement des États ? Dans les débats, on brandit souvent la menace d’une perte de confiance des marchés financiers. Je vous assure, face à l’anxiété entretenue à dessein s’affiche l’extrême sérénité de nos prêteurs. Le débat sur la dette publique n’est pas une question budgétaire, comptable et financière ; c’est un sujet hautement politique qui est donc de nature à donner lieu à débat démocratique. Le véritable enjeu, à nos yeux, est de se libérer de la tutelle des marchés financiers sur les États.

milliards d’euros, soit 112 % du PIB, avec un déficit public annoncé de 5,1 %, puis de 5,6 %, et qui pourrait finalement dépasser les 6 %, selon le Trésor. Ce dont nous discutons ici, c’est surtout du bilan, d’une vision, d’une idéologie d’un homme qui l’a incarnée pendant sept ans, Bruno Le Maire, sans oublier ses complices : les ministres

incomparable : 1 000 milliards d’euros de dette supplémentaire depuis 2017 ! Bien sûr, les soutiens du Président de la République et de l’ancien ministre ne cessent de rappeler que la période a été marquée par des crises importantes auxquelles il a fallu répondre avec de l’argent public. Ils ont raison de le rappeler,

l’économie ont été extrêmement efficaces, mais pour certains seulement. Entre 2017 et 2023, le patrimoine des cinq cents plus grandes fortunes françaises a été multiplié par deux, passant de 600 à 1 200 milliards d’euros. Notre dette a donc fait quelques heureux. Tous ces cadeaux financés par celle ci ont eu une conséquence directe dont nous mesurons aujourd’hui les effets : moins de rentrées fiscales, moins d’argent pour alimenter des services publics qui s’en trouvent dépréciés. On ne peut y voir qu’un cercle vicieux dont nous connaissons la justification idéologique : affamer

de déficit en proposant quelques timides hausses d’impôt çà et là – nous verrons à cet égard ce que nous réservera le projet de loi de finances à venir –, une bonne partie de l’effort va être fait sur le dos des ministères qui préparent l’avenir et les services publics. En définitive, on change d’équipe, on change un peu de méthode, mais on ne touche pas au fond du programme.

notamment par le biais des émissions de gaz à effet de serre. Depuis les débuts de l’ère industrielle, l’humanité a émis plus de 1 700 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Notez que 1 032 milliards de tonnes ont été émises par l’Europe et l’Amérique du Nord, soit les deux tiers du total

L’angle du climat n’est qu’une facette de la dette écologique ; il y en aurait bien d’autres. Combien d’espèces vivantes ont disparu ? Combien d’habitats ont été dégradés ou détruits, et avec eux les services écosystémiques qu’ils rendaient ? Combien de limites planétaires ont été dépassées chaque année de plus en plus tôt ? N’oublions pas que cette dette n’est pas remboursable : elle se paiera cash en vies détruites, en déplacements forcés, en souffrances multiples. L’urgence absolue est d’éviter l’emballement fatal et le chaos qui suivra. Face à l’urgence, il nous faut, nous pays occidentaux, agir et investir aujourd’hui pour la transition et l’adaptation au changement climatique. France Stratégie réévaluait hier les besoins déjà décrits l’an dernier dans le rapport de Jean Pisani Ferry

Pour cela, au lieu de sabrer ces dépenses d’avenir, il faudra trouver des financements et des recettes, mais aussi accepter de continuer parfois à s’endetter pour assurer un avenir viable. Dette budgétaire et dette écologique sont liées, mais elles ne font pas peser la même menace sur notre avenir. Toutefois, aujourd’hui, ce sont les deux faces d’un même problème, celui de l’accaparement des ressources et de la prédation des plus aisés. S’y attaquer doit être bénéfique à la fois au climat et à notre avenir : c’est la conviction profonde des écologistes depuis toujours. La parole

il peut être contre productif de les inquiéter exagérément, sauf à vouloir faire passer des mesures de redressement particulièrement impopulaires. La dette en elle même est elle un gros mot ? Les Français savaient bien que les seules familles qui s’enrichissent dans notre pays sont celles qui s’endettent. Pour un État, c’est la même chose. Il y a d’ailleurs de nombreuses bonnes raisons de s’endetter : lissage des impôts dans le temps, financement d’infrastructures, renflouement des banques,

rapport Draghi –, ou être en difficulté dans un pays faiblement endetté ? Autrement dit, faut il mourir sans dette ?

Cette dette climatique a une valeur économique calculée comme le coût des dommages engendrés par le rejet d’une tonne supplémentaire de CO2 dans l’atmosphère et, quelle que soit la définition retenue, le prix social du carbone suit une évolution exponentielle. Tout retard pris dans la décarbonation aujourd’hui sera payé plus cher par les générations futures. Dans une note de 2020, l’Insee évaluait, dans une approche comptable, le prix social du carbone à environ 500 euros en 2030, à 1 010 euros en 2040 et à 2 050 euros en 2050. 2050. À l’instar de notre trajectoire financière, celle de notre dette écologique n’est pas soutenable. Plusieurs textes engageants sont attendus : programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), nouvelle stratégie nationale bas carbone (SNBC) et plan national d’adaptation au changement climatique Malheureusement, je suis obligée de le dire, la dissolution ne porte pas la responsabilité de tous ces retards. Eh oui ! La discussion de ces textes et du prochain projet de loi de finances sera l’occasion de mettre en avant les outils à même d’infléchir notre dette écologique. Depuis la fin de la crise la fiscalité carbone est devenue un sujet tabou. Dans un rapport de 2024, la Cour des comptes, après avoir constaté que la gouvernance de la fiscalité énergétique était peu orientée autour des objectifs énergétiques et climatiques, invitait le législateur à une réflexion structurante tant pour garantir l’atteinte des objectifs environnementaux que pour préserver les grands équilibres budgétaires de l’État. L’élargissement du système européen des quotas de CO2, qui va augmenter le prix des énergies fossiles à partir de 2027 dans tout un tas de secteurs de notre économie, nous oblige à nous saisir de cette question à très brève échéance. Réduire notre dette climatique repose sur l’électrification des usages, avec pour corollaire un développement du réseau électrique et un verdissement de la production d’électricité. Les besoins d’investissement sont colossaux : je vous renvoie aux travaux de la commission d’enquête du Sénat portant

L’affaiblissement du puits de carbone forestier est aussi un signal. La capacité d’absorption du CO2 en France a été divisée par près de trois entre 2005 et 2023. Nous ne pourrons pas infléchir la trajectoire de notre dette climatique sans des politiques plus volontaristes permettant d’accroître la résilience des systèmes agricoles et forestiers. Réduire notre dette écologique nécessite un engagement financier significatif de la part de tous les acteurs. Les ménages devront réduire leur consommation d’énergie en isolant leur domicile et en adoptant des modes de transport moins carbonés. La puissance publique a aussi un rôle à jouer. Elle devra continuer à accompagner tous ceux qui ne choisissent pas leur empreinte carbone, mais la subissent. des collectivités territoriales ? Dans un rapport de mai 2024, l’inspection générale des finances (IGF) évaluait les investissements nécessaires pour réussir la transition écologique à 21 milliards d’euros par an d’ici à 2030, soit 40 % des dépenses d’équipement Ce montant est cohérent avec celui du rapport Pisani Ferry Mahfouz de 2023, qui imputait aux collectivités locales 20 milliards d’euros sur les 60 milliards annuels nécessaires à la transition écologique. Ce montant vient d’ailleurs d’être révisé dans une note de France Stratégie, rendue publique hier, qui évalue l’investissement national à 85 milliards d’euros, dont deux tiers d’investissements qui ne sont pas rentables sans intervention de la puissance publique.

Aujourd’hui, les collectivités portent déjà plus des deux tiers de l’investissement public, qu’elles financent à 80 % par de l’autofinancement. Toutefois, ce modèle de financement est mis à rude épreuve avec la hausse des charges de fonctionnement due à l’inflation et la baisse des dotations de l’État pour redresser les finances publiques. Je reprendrai à mon compte ces mots prononcés par Christophe Béchu quand il était ministre de la transition écologique : « À partir du moment où l’on fait des investissements pour l’avenir, la légitimité d’utiliser un emprunt est forte. Elle devient absolument évidente si cet emprunt vous permet de diminuer vos charges de fonctionnement ou les dépenses que vous auriez à faire plus tard. » Prenons l’exemple de l’éclairage public, qui représente près de 40 % des dépenses énergétiques de toutes les communes de France. Seulement 15 % des lampadaires publics utilisent aujourd’hui des LED, alors que cette technologie permet une économie d’énergie de 50 % par rapport à une ampoule classique. L’accroissement de la dette est traditionnellement perçu comme un signe de mauvaise gestion des deniers publics et de hausse future des impôts. La dette écologique nous oblige à changer de paradigme. La dette verte est à penser à l’aune des coûts de l’inaction climatique, largement supérieurs aux coûts de l’action. La multiplication des aléas climatiques entraîne déjà une hausse substantielle des primes d’assurance des collectivités. La loi de finances pour 2024 permet d’ailleurs à ces dernières d’isoler leur dette verte. Au delà du symbole, cet outil doit permettre d’exercer un effet de levier sur l’investissement ; il doit modifier le regard des agences de notation avec une meilleure valorisation des externalités positives de cette dette servir à recalculer la capacité de désendettement des collectivités ; il doit s’accompagner de conditions de financement de cette dette, par exemple par des prêts bonifiés. Dans un contexte budgétaire contraint, une réflexion globale doit être menée pour permettre aux collectivités d’assurer leur rôle clé dans la transition écologique. La fiscalité environnementale ne doit plus être un tabou, sans quoi nous n’arriverons jamais à faire coïncider transition écologique et justice sociale. Je nous invite donc tous ensemble, à la suite de Winston Churchill, à penser que « la responsabilité est le prix à payer

ici, reconnaître qu’au cours des dernières années, jamais la dette écologique n’a été sacrifiée sur l’autel de la dette financière. Preuve en est, les crédits ont chaque année augmenté.

À cette dette financière que nous avons longuement évoquée, il faut ajouter la dette écologique. Christine Lavarde et Thomas Dossus en ont largement parlé,

individualiser très précisément les dépenses d’investissement pour lesquelles un recours à l’emprunt peut être justifié et surtout sortir de la spirale de l’endettement issue des dépenses de fonctionnement

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce n’est un secret pour personne, l’année agricole 2023 avait été relativement favorable pour le revenu des agriculteurs de notre pays.

Comment expliquer ce paradoxe ? Il y a bien certaines circonstances : l’épidémie de maladie hémorragique épizootique (MHE) dans le Sud Ouest, les règles contre productives sur les prairies temporaires devenant prairies permanentes au bout de cinq ans dans les régions herbagères,

dans les périodes prospères, comme celle qui a précédé la Révolution française : « Un peuple qui avait supporté sans se plaindre, et comme s’il ne les sentait pas, les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s’en allège. Les économistes savent bien que la crise, ce n’est pas le point bas, mais, au contraire, le point haut ; c’est le retournement, le point de bascule. Les agriculteurs, avec leur bon sens paysan, pressentaient le retour à la réalité et les difficultés du lendemain devant lesquelles ils sont maintenant. L’année agricole qui se termine n’a pas démenti leur pressentiment : elle a été calamiteuse et a même été, sans doute, l’une des plus mauvaises depuis plusieurs décennies.

Si l’on suit l’adage de Tocqueville, après cette année moins prospère, il n’y aura peut être pas de révolte agricole cet hiver – peut être ! Mais est ce une raison valable pour oublier les revendications légitimes formulées par les agriculteurs l’hiver dernier ? Le Gouvernement peut il se permettre, l’orage passé, de remiser au grenier les engagements qu’il a pris au printemps dernier ? La réponse est non, et résolument non.

en temporisant sur le Pacte vert et en adaptant certaines bonnes conditions agroenvironnementales (BCAE), sur les prairies ou sur les jachères, ce dont nous nous sommes félicités le 9 avril dernier dans une proposition de résolution européenne du groupe de suivi de la PAC, commun aux commissions des affaires économiques et des affaires européennes du Sénat.

Or si l’on fait le décompte de ce qui n’a pas été obtenu, ou du moins pas encore, il reste beaucoup à faire. Je citerai quatre chantiers. Premièrement, les prêts garantis, que j’ai proposés dans le dernier projet de loi de finances, ne sont toujours pas devenus réalité, même si le Premier ministre les a une nouvelle fois promis, vendredi dernier, depuis le sommet de l’élevage. Dans un contexte où les taux d’intérêt sont encore élevés et où les besoins d’investissement de la ferme France sont considérables, je crois qu’il s’agit d’une mesure prioritaire pour notre agriculture. Deuxièmement, la réflexion que le Gouvernement avait lancée sur les lois Égalim est restée en suspens après la dissolution. Or plusieurs dispositifs arrivent à échéance l’année prochaine et la place des indicateurs de coûts de production n’est toujours pas définie,

Le troisième chantier est de taille. Le Premier ministre Michel Barnier a promis une « pause sur les normes ». Nous avions organisé ici, au Sénat, un débat, en février dernier, sur l’avenir de notre modèle agricole. J’avais été amené à prendre la parole et j’avais alors souligné

à nous faire cette promesse. Je voudrais là encore citer Tocqueville, qui rappelait cette évidence : « Rien n’est plus superficiel que d’attribuer la grandeur et la puissance d’un peuple au seul mécanisme de ses lois ; car, en cette matière, c’est moins la perfection de l’instrument que la force des moteurs qui fait le produit. » Le moteur de notre agriculture, en effet, c’est d’abord l’esprit d’entreprise et d’innovation de nos agriculteurs, de nos entreprises agroalimentaires et de nos coopératives. Ce ne sont pas les normes qui font pousser les choux, ce ne sont pas les normes qui font pousser les carottes, ce ne sont pas les normes qui font pousser les céréales, ce ne sont pas les normes qui nourrissent les vaches ! Bref, ce ne sont pas les normes qui remplissent l’assiette des Français.

pour adapter nos cultures au changement climatique et renforcer la résilience des chaînes alimentaires, tout en nous opposant à la brevetabilité de ces végétaux et en appelant à plus de transparence en aval.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n’est pas sans une certaine émotion que je monte aujourd’hui à la tribune du Sénat, où je m’exprime pour la première fois, en qualité de ministre de surcroît. Je veux commencer par vous remercier, cher Daniel Gremillet, des propos que vous avez tenus, sur lesquels j’aurai l’occasion de revenir.

En plaçant ce débat en tête de l’ordre du jour de la nouvelle session ordinaire après celui, essentiel, sur la dette publique, le Sénat a envoyé un signal fort au monde agricole. vous jouez encore une fois votre rôle de lanceur d’alerte reconnu par tous les professionnels agricoles. Sur la compétitivité de la ferme France, sur les limites du cadre législatif Égalim, sur le mal être des agriculteurs, sur les sujets forestiers, la Chambre haute a toujours visé juste lorsqu’il s’agissait d’alerter sur le sort des territoires et, surtout, sur celui des femmes et des hommes qui les font vivre et les façonnent. Élue de terrain, c’est avec cette méthode sénatoriale, si je puis dire, que je souhaite travailler en lien quotidien avec les élus locaux, les députés et vous mêmes. C’est un véritable pacte de travail que je vous propose aujourd’hui : l’agriculture a besoin de toutes les forces vives pour sortir de la crise. Car la crise qu’elle traverse est très profonde. J’ai été frappée de constater, en prenant mes fonctions, que la quasi totalité des filières agricoles connaissent des difficultés. En grandes cultures, la dernière récolte de blé est la pire depuis près de quatre décennies. Dans l’élevage, les risques sanitaires croissent et s’alimentent mutuellement. La production viticole souffre tant de la mutation rapide de la structure de la demande que d’aléas climatiques toujours plus fréquents. Nos industries agroalimentaires connaissent des risques de restructuration. Les problèmes sont partout. À ces difficultés s’ajoute le fait que les agriculteurs ont le sentiment que les promesses qui leur ont été faites l’hiver dernier n’ont pas encore été tenues. J’ai bien conscience de la gravité de la situation et je ne m’y résous pas. C’est pourquoi le Premier ministre et moi même avons souhaité agir immédiatement. Nous avons fait plusieurs annonces, au sommet de l’élevage, sur la fièvre catarrhale ovine et je suis sûre que nous en reparlerons au cours de ce débat. Des garanties ont, en outre, été apportées pour accélérer l’indemnisation des pertes des éleveurs liées à d’autres maladies vectorielles, comme la maladie hémorragique épizootique. S’agissant de la viticulture, dans la lignée de mon prédécesseur, j’ai obtenu que l’Union européenne valide un dispositif d’arrachage définitif pour un montant de 120 millions d’euros. C’était une demande majeure des filières et je crois qu’il faut s’en féliciter.

Et je veillerai à ce que, lors de nos débats sur le projet de loi de finances dans les prochains jours, les engagements fiscaux et sociaux pris par le Gouvernement l’hiver dernier soient tenus. Le monde rural nous regarde et ses attentes sont grandes. Je serai donc au rendez vous. Ces actions sont des urgences vitales, qui permettront de répondre à la crise agricole. étant, sortir l’agriculture de la crise, c’est aussi lui donner un objectif clair, un cap, une vision sans laquelle nous ne pourrons motiver les jeunes et leur donner envie de s’engager dans les métiers agricoles.

est celui du renouvellement des générations en agriculture, comme M. le sénateur Gremillet l’a rappelé. Avec près d’un agriculteur sur deux âgé de plus de 55 ans, le renouvellement n’est pas assuré et le nombre d’exploitations, qui baisse de façon dramatique depuis vingt ans, continue de décroître.

Nous réfléchissons actuellement avec la secrétaire d’État chargée de la consommation, l’une de vos anciennes collègues, Laurence Garnier, à la meilleure façon de poursuivre notre travail à vos côtés sur ce sujet.

l’agriculteur passe plus de temps dans les champs que derrière un ordinateur. Or la plupart des agriculteurs croulent aujourd’hui sous les démarches administratives. Comme l’a déclaré le Premier ministre, l’heure est à la pause sur les normes. Il faut également redonner du bon sens à la réglementation : comment expliquer à un agriculteur qu’il ne peut pas engager des travaux d’épandage, car il a dépassé la date fixée dans un texte pris à Paris, alors qu’il ne cesse de pleuvoir depuis plusieurs semaines ? C’est un point sur lequel le Premier ministre est revenu à ma demande, ce dont je le remercie.

Je veux le dire clairement à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs : l’agriculture représente un intérêt général majeur. Oui, il est primordial de rappeler que la souveraineté agricole et alimentaire de la Nation contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux,

Aux côtés des rapporteurs du texte, Laurent Duplomb et Franck Menonville, je sais d’emblée que les travaux seront ancrés dans la réalité du terrain. J’en profite pour saluer aussi la qualité des travaux conduits par les rapporteurs pour l’Assemblée nationale. Bien sûr, ce texte n’est pas suffisant. Il pourra être complété par d’autres textes, le cas échéant sur votre proposition – je suis prête à y travailler avec vous. Nous devrons ensuite répondre ensemble aux défis du temps long. Face au réchauffement climatique, nous devons dès aujourd’hui penser l’agriculture de demain avec nos voisins européens. En matière de souveraineté alimentaire, les chiffres sont très

Nous ne devons jamais transiger avec la protection de nos filières. Il y va de notre souveraineté. Aussi faudra t il lutter contre les nombreuses distorsions de concurrence dont souffrent Je soutiendrai à ce titre le projet européen d’instituer des clauses miroirs envers les États tiers qui choisissent le dumping. Nous aurons besoin pour cela d’une action internationale résolue et ferme, ainsi que du soutien de nos partenaires européens.

comme l’ont très bien compris et, du reste, écrit mes excellents collègues Laurent Duplomb et Sophie Primas dans leurs rapports sur la compétitivité de la ferme France. Fiscalité, main d’œuvre et surréglementation doivent être adaptées ; à défaut, il faudra augmenter les aides directes européennes.

signer un accord d’association avec le Mercosur en fin d’année. Madame la ministre, la France aurait elle changé de position depuis les annonces du Président de la République et les engagements du Premier ministre en début d’année ? Allez vous enfin renverser la table et sauver la souveraineté agricole ?

Un accord de libre échange est en cours de négociation : il intégrera notamment les exigences sanitaires. Il n’y aura pas de réouverture du marché européen sans l’application des standards continentaux, et ce pour éviter toute concurrence déloyale. Cette expérience doit nous inciter à faire de l’origine

M. Jean Claude Anglars. Madame la ministre, comme l’a dit Daniel Gremillet, la rentrée agricole se fait sous haute tension. La situation sanitaire, le projet de loi d’orientation agricole, le système assurantiel, le prix du fermage, l’attractivité du métier, le renouvellement des générations la liste des sujets d’actualité s’allonge, tandis que les mobilisations du monde agricole datent d’il y a plus de huit mois. Il n’y a plus de temps à perdre pour sortir de cette crise. Sans amélioration notable et rapide, notamment en ce qui concerne la rémunération des agriculteurs, au sujet de laquelle les annonces du précédent gouvernement n’ont pas eu les effets escomptés,

En Aveyron, entre 300 et 400 exploitations sont concernées. Il est urgent de faire le nécessaire pour que les délais de paiement – lequel paiement intervient habituellement à la mi octobre – soient respectés cette année. je souhaite réaffirmer la nécessaire ambition agricole de la France : la crise a révélé combien les contraintes handicapaient l’agriculture, tandis que les agriculteurs souffrent d’un manque de vision stratégique. La souveraineté alimentaire et la compétitivité sont désormais en jeu.

Vous évoquez un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l’activité agricole. C’est une évidence : il faut avoir fréquenté les agriculteurs pour savoir à quel point l’exercice de leur métier est devenu très compliqué.

le ZAN, un sujet cher à cette maison et au sénateur Longeot, qui a traité de cette question dans le cadre

Nous serons confrontés à une forte diminution du nombre de naissances d’agneaux. Par conséquent, il faudra deux, voire trois ans pour reconstituer les cheptels, si tant est que les éleveurs puissent le faire.

maladie détectée récemment qui touche, selon les chiffres fournis par votre ministère, 4 644 foyers. Par ailleurs, vous avez annoncé, d’une part, la commande par l’État de 11,7 millions de doses

permettre de mieux lutter contre la propagation de l’épizootie, pourriez vous apporter des précisions sur la mise en œuvre et le calendrier de ces mesures, ainsi que sur la prise en compte du remboursement des vaccins s’agissant de la FCO de sérotype 8 ?

qui constituent des revenus importants pour les agriculteurs et dont le montant ou l’ampleur est très souvent lié au nombre d’agneaux vendus. Dans un contexte où l’agriculture traverse une crise majeure et où la prédation sévit dans de nombreux territoires, les prêts garantis par l’État (PGE) pourront ils être accordés aux éleveurs, afin de les aider à reconstituer leurs cheptels ? enfin de prévoir un retour d’expérience pour tirer les enseignements de cette crise catastrophique et éviter de reproduire certains dysfonctionnements constatés – équarrissage, distribution des vaccins, retard des laboratoires d’analyse –, tout en mettant en place le soutien psychologique que les éleveurs

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelle agriculture voulons nous pour demain ? Derrière cette question fondamentale qui englobe tous les enjeux, qu’ils soient environnementaux, économiques, fonciers ou de santé publique, il y a la problématique du renouvellement des générations et de l’attractivité du métier. Quand les tracteurs ont quitté les champs en signe de colère pour signifier le mal être des paysans, les Français ont découvert une profession en danger. La lourdeur administrative met en péril la santé des entreprises et vient affaiblir notre compétitivité sur un marché où la concurrence internationale est exacerbée.

Les agriculteurs l’ont dit et redit en janvier dernier : ils sont à bout de forces, à bout de souffle ! Ils souffrent de problèmes de revenus que nous n’avons pas le droit de nier. Je citerai quelques exemples : les prédations et les épidémies qui se développent affaiblissent les éleveurs

pour les bénéfices qu’ils offrent à la société : restructuration des sols qui captent le dioxyde de carbone, lutte contre les incendies, préservation des écosystèmes, façonnage des paysages. Ma question est donc simple, madame la ministre : avez vous prévu des mesures en ce sens dans la future LOA, qui

Je suis très favorable au principe d’une meilleure valorisation des externalités positives de l’agriculture. Il y en a beaucoup : le stockage du carbone dans les sols, la biodiversité, l’aménagement du territoire en sont quelques exemples.

engagement en faveur d’une ruralité qui ne veut pas baisser les bras. C’est la ruralité que je connais, que j’aime et que je veux défendre.

la propagation fulgurante de la fièvre catarrhale ovine est un nouveau coup dur pour nos agriculteurs, qui font déjà face à des difficultés économiques notamment causées par des conditions météorologiques

Les éleveurs se sentent démunis face au manque d’anticipation au niveau tant européen que national, et face à une réponse trop tardive. À cet égard, les réponses apportées par le Gouvernement lors du sommet de l’élevage vont dans le bon sens. Nos agriculteurs doivent être soutenus et accompagnés, non seulement pour faire face aux surcoûts en matière sanitaire, mais aussi pour reconstituer leurs cheptels décimés. Madame la ministre, pourriez vous préciser les mesures que vous comptez mettre en œuvre, et dans quels délais ? Quels enseignements tirez vous de cette crise et de ce manque de coordination européenne dans la prévention comme dans les stratégies vaccinales suivies ? Comment expliquer le retard de la réponse vaccinale française face à une maladie pourtant bien connue et à la vitesse de propagation fulgurante ? La parole est à Mme la ministre. Monsieur le

la production viticole pourrait être inférieure de 10 % à 16 % par rapport à l’année 2023, et même de 30 % dans le Gard. Quant aux éleveurs, ils font face à trois épizooties en même temps,

Enfin, l’objectif d’autonomie alimentaire est essentiel pour garantir notre souveraineté alimentaire, et pour cela il nous faut donner la priorité à l’approvisionnement des populations par des productions locales.

en renforçant le sentiment d’abandon du monde paysan et agricole.

d’euros. des marges que Lactalis réalise sur les différents segments du marché laitier ? de la poursuite des importations de lait par Lactalis en France ? Quel déplorable message envoyé, alors que les agriculteurs se battent tous les jours pour redynamiser le secteur et que la filière appelle au renouvellement des générations !

Où est l’humain dans cette affaire ? Ce scandale démontre un peu plus, s’il le fallait, l’urgence qu’il y a à remettre en place une régulation publique des marchés. Pour garantir des prix rémunérateurs et une répartition des volumes dans les bassins laitiers, il faut instaurer une régulation publique des volumes, et mettre fin à cette dérégulation à la main des industriels et dictée par leur seule soif de profit. Car oui, cette stratégie de Lactalis vise à mettre au pas les éleveurs laitiers français. Voilà le monde merveilleux du marché mondialisé et de sa compétitivité, si chers à certains dans une recherche effrénée du moins disant social et environnemental, et du mieux disant fiscal ! Madame la ministre, apporterez vous une réponse politique à la stratégie mortifère de ces industriels, qui met à mal notre souveraineté agricole et nos paysans ? Engagerez vous des réformes structurelles pour établir enfin des règles justes et équitables dans les relations commerciales

la viticulture est victime du changement climatique – gel, grêle, sécheresse à répétition – et d’un marché atone. Sur le terrain, dans l’Aude, on me dit tous les jours : « Dites leur, à Paris, ce qui se passe ! Aidez nous ! » Alors, écoutons les Ludovic a les mots justes lorsqu’il dit que « l’arrachage sera le plus grand plan social dans l’histoire du Languedoc ». Frédéric ne veut pas être celui qui mettra fin à l’histoire de générations entières de vignerons. Mais si certains, comme lui, vont les plus jeunes. Ainsi, Maxime et Émilie veulent « faire évoluer leur exploitation pour la rendre compétitive ». Mais comment investir en période de crise ? Écoutons Amandine nous dire : « Avec l’inflation, tout augmente, sauf le prix du vin Comment payer nos charges et nos emprunts ? » Il est urgent de restructurer la dette bancaire de la filière. Écoutons Lilian nous dire : « Ma coopérative fait une demi récolte ; on utilise la moitié de notre outil de production, alors pourquoi l’amortit on à taux plein ? » Madame la ministre, le destin climatique de la France se joue chez nous, dans l’Aude et les Pyrénées Orientales. C’est pourquoi votre politique agricole doit prévoir une exception méditerranéenne, dotée de moyens à la hauteur. Ainsi, Jean Marie a raison de demander « un fond de transformation de la filière ». Il convient bien sûr de répondre à la question de l’eau, non pas pour surproduire, mais pour sécuriser la production. Actuellement, il pleut moins à Leucate qu’au Sahara ! Comme le disent si bien Roland et Annie : « Sans eau, il n’y a pas de vigne ; sans eau, il n’y a pas de vie. » Sans eau, il est vain de parler de cultures alternatives. Écoutons encore Philippe nous Je ne produis pas seulement du vin, je protège les paysages. La vigne est plus efficace que les Canadairs pour lutter contre les incendies ; elle est d’utilité publique. » Quant à Gérard, il peine à promouvoir ses vins sur le marché mondial les réseaux sociaux, comme le font ses concurrents américains, à cause d’une loi Évin inadaptée à la révolution numérique. La viticulture vacille. Je ne peux me résigner à voir la vigne disparaître sans agir. La filière ne doit pas subir le sort de la sidérurgie. Attention, ce que nous ne produirons plus en France sera produit par d’autres, ailleurs Ne laissons pas nos territoires être doublement désertés, par le climat et par la République. Madame la ministre, Sebastien, vigneron et sénateur, vous lance une invitation solennelle : venez dans l’Aude constater par vous même l’ampleur de la crise et écouter Ludovic, Philippe, Émilie, Gérard et tous les autres ! La parole est à Mme la ministre.

où la France sera la puissance invitante de tous les pays de l’Union européenne, tandis que, dans le même temps, la viticulture vit un drame. C’est particulièrement le cas dans votre département, où le déficit en eau est dramatique.

à notre balance commerciale et crée des milliers d’emplois, se trouve dans une situation très critique. En janvier dernier, la Chine lançait une enquête antidumping menaçant gravement nos exportations de cognac et d’armagnac.

que les autorités chinoises imposeront dès le 11 octobre des droits additionnels de 35 % sur les spiritueux européens, notamment le cognac et l’armagnac.

La filière, qui a le sentiment d’être sacrifiée, avait pourtant averti que ce vote risquait d’entraîner des rétorsions sur nos spiritueux. Elle demande donc qu’une solution soit négociée pour écarter toute surtaxe sur nos produits en Chine, de manière que chaque partie sorte par le haut de cette situation de blocage. C’est urgent, madame la ministre ! Le 17 septembre, à la veille des vendanges, une manifestation avait mobilisé de nombreux participants. Attendez vous à de très fortes mobilisations dans nos territoires si rien n’est fait.

modèle du pacte Dutreil ; l’application du principe « pas d’interdiction sans solution » pour les produits phytosanitaires ;… Bravo ! … la révision de la moyenne olympique pour l’assurance climatique ; le maintien d’une fiscalité qui permette une consommation modérée, mais accessible, de nos produits

Enfin, nous continuons de travailler avec l’Union européenne sur l’approbation des clauses miroirs, dont vous connaissez bien le principe, pour protéger à la fois les consommateurs et les producteurs. Pour ce faire, nous avons recueilli l’accord et le soutien de l’Allemagne, des Pays Bas, de l’Autriche et de l’Irlande. Il est très important que la France ne soit pas isolée. C’est la raison pour laquelle nous avons fait adopter un protocole annexe à l’accord, qui bloque l’accord avec le Mercosur. Nous ne pouvons pas laisser entrer en France 99 000 tonnes de bœuf, 100 000 tonnes de volailles, 180 000 tonnes de sucre

Le peu de jeunes agriculteurs qui s’installent en ce moment seront encore en activité en 2050. Autrement dit, si nous n’intégrons pas cette donnée climatique dans la manière dont nous pensons et accompagnons notre agriculture, nous nous dirigeons tout droit vers une catastrophe. Le Premier ministre a annoncé une grande conférence nationale sur l’eau. Sans eau, il n’y a pas d’agriculture. Sans eau, il n’y aura pas d’agriculteurs. Il est donc essentiel que cette conférence associe tous les acteurs, y compris le monde agricole, afin de définir une stratégie globale pour assurer un usage raisonné de l’eau et un juste partage de cette ressource. Cette stratégie nationale devra ensuite se décliner localement à l’échelle des bassins versants. Madame la ministre, mon département connaît aussi bien la sécheresse que les inondations. Sur des territoires comme celui ci, des solutions doivent être rapidement trouvées pour stocker l’eau, lorsqu’elle est excédentaire, avant qu’elle ne parte à la mer. parte à la mer. Le dérèglement climatique implique également une multiplication de l’ensemble des aléas. Les pertes de récoltes sont non plus l’exception, mais la règle. Dans ce contexte, la référence olympique fait perdre toute attractivité à l’assurance récolte. Il est urgent de discuter avec l’OMC d’une révision de ce référentiel. Mon territoire est particulièrement exposé à ces difficultés. De plus, notre modèle agricole méditerranéen fragilise cette agriculture, qui est pourtant axée vers la qualité.

du changement climatique en cours sont particulièrement visibles sur nos ressources en eau, avec des sécheresses plus importantes l’été et, vous l’avez également souligné, de fortes précipitations. D’où l’idée que, quand l’eau est abondante, on puisse la capter,

Les conditions climatiques extrêmes ont entraîné des rendements historiquement bas pour nos agriculteurs, déjà grandement fragilisés par l’inflation et pressurés par la surtransposition des normes.

conséquences pour l’écosystème céréalier, puisque la baisse des volumes fragilise le financement des instituts, notamment Arvalis, et ralentit les actions collectives de

mettra en péril notre souveraineté et notre commerce alimentaire, dans un contexte géopolitique incertain.

Tout d’abord, pour les grandes cultures, le déclenchement de l’assurance récolte garantira que tous les exploitants touchés de manière exceptionnelle bénéficient d’une indemnisation. Je rappelle que, jusqu’à la réforme de 2023, les grandes cultures ne bénéficiaient pas du régime des calamités agricoles. Ensuite a été mis en place

de soutien que je trouve intéressant : il s’agirait d’octroyer des prêts bancaires adossés à une garantie d’État, afin de permettre de passer cette période difficile.

Avec plus de 4 600 foyers touchés, la FCO et la MHE continuent de s’étendre inexorablement et affectent non seulement les ovins, mais encore les bovins et les caprins sur l’ensemble du territoire. Face à cette menace, les mesures gouvernementales restent largement insuffisantes. Le fonds de 75 millions d’euros que vous avez alloué pour la FCO

du mois de juin prochain. Comment tolérer une telle situation ? Cette crise dépasse la seule question des compensations économiques. Sans doute, nous devons commencer par indemniser au juste niveau chaque bête perdue, chaque agneau, chaque chevreau

quotidien qui les conduisent tout droit vers une détresse psychologique alarmante. Un soutien psychologique est indispensable. Ignorer cet aspect, c’est condamner nos éleveurs à l’épuisement mental et même parfois, malheureusement, au pire. Madame la ministre, il ne s’agit plus d’utiliser des rustines : nos éleveurs exigent des réponses concrètes et des solutions durables ! Le moment est venu de réviser en profondeur le plan loup, d’y apporter des ajustements répondant réellement aux attentes des éleveurs tout en tenant compte des impératifs environnementaux.

Vous le savez, la prédation du loup est un véritable fléau pour le pastoralisme, et il faut continuer d’agir en faveur de nos éleveurs. Nous avons donc tous accueilli avec satisfaction la récente décision de l’Union européenne d’abaisser le statut de protection du loup. Toutefois, il reste encore au comité permanent de la convention de Berne à adopter cette mesure, et à la directive dite Habitats faune flore du 21 mai 1992 d’être amendée en conséquence. Madame la ministre, êtes vous confiante dans l’avenir de cette décision à l’échelon européen et que mettez vous en œuvre pour qu’elle aboutisse ?

en œuvre une expérimentation pour la protection des troupeaux de bovins, lesquels ne peuvent faire l’objet de la même protection que les ovins, avec la possibilité d’un tir de défense simple lorsque la présence d’un loup est constatée. demande en faveur de la généralisation de cette solution, qui s’avère très efficace face à l’augmentation significative du nombre de bovins prédatés

Est ce une mesure que le Gouvernement serait prêt à généraliser rapidement ? Pour conclure, je souhaite aborder la question des indemnisations. Vous avez mentionné, madame la ministre, les compensations des pertes directes liées à la prédation du loup, mais qu’en est il des pertes indirectes ? Celles ci ne sont pas suffisamment valorisées,

est à Mme la ministre. Madame la sénatrice Martine Berthet, vous évoquez un sujet sur lequel j’ai moi même beaucoup travaillé. En effet, une étape importante a été franchie à Bruxelles

En effet, six mois après les vives tensions qui ont secoué le monde agricole dans le pays, plus particulièrement dans le Lot et Garonne, je souhaite vous faire part de ma vive inquiétude

du revenu des agriculteurs, des normes et de la réglementation, auxquels se sont ajoutés au cours des six derniers mois les problèmes climatiques affectant le blé, le soja, le maïs, le sorgho,

La profession agricole a le sentiment d’être délaissée. Elle estime ne pas être écoutée et se demande si son activité a encore du sens. La colère

Madame la ministre, je sais que ce sujet vous préoccupe ; c’est la raison pour laquelle je vous demande de nous apporter des précisions pour répondre à cette colère annoncée. est à Mme la ministre. Madame la sénatrice Christine Bonfanti Dossat, je sais votre extrême vigilance sur ces questions. Vous m’avez alertée à ce sujet, et je vous en remercie parce que le regard des parlementaires, bons connaisseurs de leur territoire,

le retard dans la mise en œuvre des annonces de mon prédécesseur, l’aggravation de la crise climatique, avec des sécheresses importantes

Mais ces excès sont à la mesure de l’inquiétude ressentie : ces métiers ne veulent pas disparaître, ces agriculteurs aspirent à vivre de leur métier sur le territoire qu’ils aiment, où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils travaillent.

avec la mort des animaux, mais aussi des pertes indirectes, avec des avortements, une baisse de la production laitière, voire des problèmes de fertilité. Les éleveurs peinent donc à exporter leurs animaux vers des pays

Aussi, face à la menace croisée de la fièvre catarrhale de sérotypes 3, 4 et 8, et de la maladie hémorragique épizootique, les éleveurs demandent la gratuité des vaccins pour l’ensemble des maladies vectorielles. À l’échelle nationale, plus de 3 800 foyers de contamination sont recensés.

je comprends très bien que plusieurs de vos collègues aient choisi de l’évoquer. Les enjeux sont bien d’accompagner les élevages atteints et de lever les blocages qui peuvent exister, notamment en matière d’exportations.

travailler sur cette question à l’échelon européen, car on sera toujours en retard d’un vaccin. C’est la raison pour laquelle mon prédécesseur avait évoqué l’idée d’une banque d’antigènes

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un spectre hante la France agricole ! Ce spectre, c’est celui de la décapitalisation, notamment de notre cheptel bovin et ovin, durement touché par des crises sanitaires qui n’existent pas depuis hier, mais qui s’amplifient. Ce spectre, c’est celui du déclin de notre compétitivité et de la perte de marchés, notamment au sein du marché intérieur avec nos concurrents européens directs. J’avais annoncé en 2019 que nous connaîtrions une balance commerciale déficitaire ; nous y sommes Ce spectre, c’est également celui de l’érosion de notre souveraineté alimentaire, voire celui de menaces pour notre sécurité alimentaire, si les tendances à l’œuvre se poursuivent. En un mot,

! Cette liquidation est le fruit de la Sainte Alliance d’une technocratie abrutissante et des dogmes environnementaux. J’ai écouté tous mes collègues, et je vous ai écoutée attentivement, madame la ministre, comme je l’avais fait la semaine dernière lors du sommet de l’élevage.

d’autant que ce texte avait été enrichi d’un volet de souveraineté et d’un volet de simplification des normes environnementales, qui vont dans le bon sens.

Sur le terrain, les agriculteurs attendent dès maintenant le desserrement de l’étau normatif et ils veulent que nous les sortions des impasses techniques dans lesquelles nous les avons mis malgré eux, année après année. À cette fin, j’ai proposé une méthode pour sortir plus efficacement de cette crise. Cette méthode consiste à saucissonner et à conditionner. Elle s’articule en quatre temps.

faut un texte législatif au format réduit, concentré sur les principales entraves aux activités agricoles, qui serait déposé en octobre ou en novembre, pour redonner de la souplesse en matière d’usages de l’eau

Quatrièmement, en parallèle, et dès aujourd’hui, je vous propose, madame la ministre, d’avancer sur des mesures de simplification par voie réglementaire

budget, entraves, LOA : voilà ma proposition, madame la ministre. Êtes vous prête à nous suivre dans cette direction ? Les agriculteurs vous attendent et nous attendent : il s’agit de les sortir du mauvais pas dans lequel vos prédécesseurs les ont mis.

exemple : « Cet État se veut si bienveillant envers ses citoyens qu’il entend se substituer à eux dans l’organisation de leur propre vie. Ira t il jusqu’à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d’eux mêmes ? […] Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui. » Je peux vous le dire, les agriculteurs méditent Tocqueville

Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur, pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour d’un droit de réplique, pour une minute. Madame la ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui ci aura retrouvé sa place dans l’hémicycle. Dans le débat,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, trouver un rendez vous chez un généraliste, un spécialiste, un kiné ou un psy est devenu en France une galère quotidienne. On nous en parle tous les jours et nos concitoyens comme les élus locaux sont démunis face à la défaillance de l’offre de soins. La récente mission d’information du Sénat sur la santé périnatale a aussi démontré le déficit de gynéco obstétriciens, d’anesthésistes, de pédiatres, de sages femmes.

La situation des urgences commande aussi une telle réponse. De plus en plus de nos services ferment de manière intermittente, comme à Lillebonne ou à Fécamp, dans mon département, où la pression s’accroît sur le groupe hospitalier du Havre, dont les agents sont mobilisés depuis onze semaines pour alerter sur cette situation intenable. Des gouvernements successifs ont instauré et maintenu, depuis les années 1970, le dans les études de santé, ce qui a fait chuter le nombre d’étudiants en médecine de 8 500 en 1971 à 3 500 en 1990. L’objectif était de réduire les dépenses de santé. Chacun le reconnaît aujourd’hui, cette solution austéritaire s’avère une bombe à retardement. La population a en effet augmenté et vieilli ; et les professionnels de santé aspirant légitimement à conjuguer vie professionnelle et vie privée, le nombre de médecins comme le temps médical disponible ont diminué à mesure que les besoins s’accroissaient. Le a été supprimé en 2021 et nous avons salué cette suppression. Mais la réforme des études de santé, mise en œuvre à la rentrée universitaire 2020 2021 de manière particulièrement chaotique, a laissé sur le carreau des centaines d’étudiants qui se destinaient à être médecins : un vrai gâchis

qui nous conduit à penser qu’il faut supprimer le, financer l’augmentation des capacités de formation des universités et développer les terrains de stage. La faculté de médecine de Rouen, par exemple, a augmenté ses capacités d’accueil de plus de 200 % en vingt ans, à moyens quasi constants. Comment faire plus sans enseignants, sans bâtiments, sans services universitaires supplémentaires ? Il faut former davantage, mais aussi former mieux. Nous ne pouvons accepter que les internes continuent de pallier les pénuries de médecins en travaillant les nuits et les week ends pour seulement 6 euros de l’heure Dans son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière que « la lutte contre les déserts médicaux et contre la pénurie de soignants sera[it] l’une des priorités de [s]on gouvernement. Le temps est révolu, a t il poursuivi, où l’on avait la crainte de former trop de médecins. Nous allons amplifier l’effort engagé. » Nous disons : « chiche ! », même si l’annonce d’une diminution drastique de la dépense publique est contradictoire avec cet objectif. Et nous proposons, comme le font des collègues venant de différentes familles politiques,

Il montre aussi que ce frémissement ne comble pas les inégalités territoriales ; au contraire, celles ci se creusent. Un département comme l’Eure, par exemple, dispose de moins de 80 médecins pour 100 000 habitants, soit moitié moins que dans les départements qui comptent de grandes métropoles. L’absence de professionnels de santé en nombre suffisant fait peser sur les épaules des internes et des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) le maintien des services hospitaliers. Les Padhue sont en première ligne dans les services des hôpitaux désertés

pour garantir aux Padhue des conditions dignes de travail et de vie. Le « programme Hippocrate » annoncé par le Premier ministre, dans le cadre duquel internes français et étrangers s’engageraient volontairement à exercer dans les territoires qui manquent le plus de médecins, ne devra pas être hypocrite. Les collectivités n’ont pas attendu pour financer les dépenses de transport ou de logement d’étudiants venant en stage dans leur territoire, ni même pour financer des postes de chefs de clinique dans les universités, même qu’elles multiplient par ailleurs les mesures pour accompagner les professionnels qui viennent s’installer. Elles ne pourront pas assumer indéfiniment cette charge seules. Surtout – on y revient toujours –, il faut former des médecins pour qu’ils viennent exercer dans tous les territoires. et des statistiques (Drees) parue au mois de juin dernier, les médecins des zones rurales ont ou vécu pendant leur enfance en zone rurale, ou effectué au moins un stage en zone rurale, ou effectué des remplacements d’au moins trois mois en zone rurale. En France, depuis quelques années, plusieurs facultés de médecine proposent de décentraliser les enseignements de la première année des études de santé vers des villes moyennes – je pense à Pontivy, rattachée à la faculté de médecine de Rennes, ou à Périgueux, rattachée à Bordeaux. Le déploiement des stages universitaires des étudiants en médecine dans les territoires ruraux doit encore être renforcé ; c’est la condition pour former davantage et c’est aussi un facteur avéré d’installation future en zone rurale. rurale. Aussi est il à nos yeux nécessaire de démocratiser les études de santé, car, au risque d’être un peu caricaturale, j’affirme que plus il y aura de jeunes médecins issus des quartiers populaires ou des zones rurales, moins les médecins verront d’obstacles à s’y installer. Il y a donc aussi

figure parmi les premières préoccupations de nos concitoyens : ceux ci ne sauraient admettre que, dans un pays comme la France, en 2024, l’on ne puisse pas avoir accès à un médecin quand c’est nécessaire. Je remercie d’avance chacune et chacun de sa contribution à ce débat.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans nombre de territoires, il suffit d’essayer de prendre rendez vous avec un médecin, généraliste ou spécialiste, ou bien d’aller aux urgences pour rapidement parvenir à un constat évident : notre pays manque de médecins. Je m’en excuse d’emblée auprès des soignants : mon intervention traitera davantage des médecins que des soignants au sens large, car je pense que « la nécessité de former davantage de médecins » soulève en elle même beaucoup de questions, et ce traiter le sujet de l’accès aux soins nécessite, en pratique, de se pencher sur la question de la coopération entre tous les professionnels de santé. En 2024, le nombre de médecins, y compris remplaçants et retraités actifs, est d’environ 237 000, contre 215 000 il y a à peine quinze C’est donc 22 000 de plus, et cette augmentation est tout aussi encourageante que frustrante : comment peut on ne pas réussir à faire mieux avec plus ? Tout d’abord, il est évident que les nouveaux médecins travaillent différemment par rapport à ceux des générations précédentes. Beaucoup d’entre eux, et c’est bien légitime, recherchent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ne souhaitent plus travailler douze heures par jour six jours – voire Ensuite, plusieurs facteurs concourent à ce que les besoins de la population en matière de soins augmentent : le vieillissement de la population, l’augmentation de la dépendance, l’explosion des maladies chroniques ou encore la dégradation de la santé mentale. est donc nécessaire de continuer à former davantage de médecins et, plus largement, de soignants. Mais il est tout aussi nécessaire d’optimiser le temps médical que représentent ces effectifs supplémentaires. Les difficultés sont connues depuis longtemps. évidemment commencer mon propos sans mentionner le problème de la surcharge administrative : un accident du travail, par exemple, implique la rédaction d’un certificat médical initial, éventuellement d’un arrêt de travail, d’une ordonnance, d’une feuille de soins, etc.

L’informatique représente aussi une perte de temps ahurissante. Comment est il possible que, dans certains – je dis bien « certains » – hôpitaux, en 2024, il n’y ait pas de logiciel unique ? Un médecin doit se connecter sur le logiciel des scanners, puis, un mot de passe différent, sur le logiciel de biologie, et ainsi de suite en fonction des examens nécessaires. Un urgentiste me disait récemment : « Cinq minutes avec un patient, c’est quinze minutes d’informatique. aussi le problème de la répartition des médecins sur le territoire et parmi les différentes spécialités ; la psychiatrie, et notamment la pédopsychiatrie, est en grande souffrance. J’en profite d’ailleurs pour saluer le choix du Premier ministre de faire de la santé mentale la grande cause nationale de 2025.

Optimiser le temps médical, cela relève aussi de la responsabilité des patients. Il est tout bonnement inacceptable qu’un patient se rende aux urgences parce qu’il a le nez qui coule, qu’il bénéficie d’un examen et d’un traitement qui doit durer quatre jours et qu’il retourne aux urgences le lendemain… car il présente exactement le même symptôme. Heureusement, un tel cas ne représente pas la majorité des patients ; mais il y a là une réalité dont tous les médecins vous parleront. Responsabiliser, cela ne veut pas dire pénaliser les plus démunis : cela veut dire sanctionner les abus – et c’est une nécessité.

automatiser l’usage du dossier médical partagé (DMP), alléger et simplifier la charge administrative. Madame la ministre, ma question est plutôt simple

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier nos collègues du groupe CRCE – Kanaky d’avoir demandé l’inscription à l’ordre du jour de notre assemblée de ce débat sur la nécessité de former davantage de médecins et de soignants,

! Oui, madame la ministre, il faut former plus de médecins et de soignants dans notre pays, pour l’hôpital comme pour la ville ! L’affirmation est simple, et la réponse attendue rapidement sur le terrain, voire urgemment dans certains territoires, alors que le sujet de la formation s’inscrit dans un temps long.

Et je salue les propos qu’il a tenus lors de sa déclaration de politique générale, qui ont déjà été rappelés : « Le temps est révolu où l’on avait la crainte de former trop de médecins. » Je m’en réjouis d’autant plus que le groupe Les Républicains a proposé dans son pacte législatif, avant la constitution du Gouvernement, une loi santé dont les grands axes sont clairement énoncés.

Je parlerai essentiellement de médecine générale, pierre angulaire de notre système de santé en ville. Former davantage de médecins, c’est territorialiser les études de médecine. C’est continuer à créer des antennes universitaires de première et deuxième années d’études, parfois plus accessibles pour les étudiants, tant géographiquement que financièrement. C’est revoir la réforme récente de la première année d’études de santé : il n’est pas acceptable que la réforme dite Pass (parcours accès santé spécifique) – LAS (licence accès santé) ne soit pas appliquée de la même manière dans toutes les universités. Certaines universités ont même inventé la « LAS 50 50 » ; je vous laisse y réfléchir…

évolution souhaitée par le Sénat le vote de la proposition de loi de Bruno Retailleau avant d’être introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il conviendra surtout, madame la ministre, de veiller Il conviendra surtout, madame la ministre, de veiller à ce que les stages afférents soient prioritairement réalisés en ambulatoire dans des zones sous denses, plutôt qu’orientés vers l’hôpital par dérogation. Bien sûr, il faudra en contrepartie que la qualité de l’accueil réservé à ces futurs médecins soit au rendez vous, sur le plan tant des locaux que de l’accompagnement professionnel.

Former plus, c’est aussi corriger les effets négatifs de la réforme des études de santé, laquelle a affecté, par exemple, la filière pharmacie – ma collègue l’a rappelé. Depuis la réforme, cette filière n’est plus visible et les deuxièmes années de pharmacie ne font plus le plein

Madame la ministre, mes questions sont simples. Comment pensez vous vous saisir des propositions faites par le groupe Les Républicains du Sénat en matière de santé ? Comment envisagez vous de travailler avec votre collègue ministre chargé de l’enseignement supérieur pour corriger la réforme des études de santé ?

Nous attendons ses conclusions, qui ne devraient pas tarder. Bien qu’il soit trop tôt pour estimer les effets à long terme de cette réforme, il sera sans doute opportun de réfléchir à des ajustements.

semble donc que je vais signer des décrets très rapidement…

La préoccupation de l’accès à des soins de qualité pour tous, partout sur notre territoire et à tout moment de la vie, nous rassemble sur toutes les travées. Je ne l’apprends à personne, la France fait face à une pénurie croissante de soignants et de médecins, avec des déserts médicaux dans de nombreuses régions. On estime aujourd’hui que près d’un Français sur trois vit dans un désert médical. Par ailleurs, le vieillissement des médecins et de la population exige une augmentation de l’offre de soins. Nous le voyons tous dans nos territoires respectifs : nos hôpitaux, nos Ehpad, nos centres de soins et nos cabinets libéraux sont sous tension permanente. Partout en France, des postes restent vacants, les services d’urgence saturent et les listes d’attente pour consulter un spécialiste s’allongent. La solution la plus évidente pour remédier à ces pénuries, révélées notamment par la crise sanitaire, est d’augmenter le nombre de praticiens en formant davantage. C’est un impératif pour l’avenir. Pour les médecins, le a été supprimé en 2020, sous l’impulsion du Président de la République. Quatre ans après cette réforme si nécessaire, nous en constatons déjà les premiers résultats. On observe une nette augmentation du nombre d’étudiants accédant à la deuxième année de médecine. De 8 150 en 2017, le nombre de places en médecine à l’université est passé à 10 000 en 2023. Il augmentera à 12 000 places par an en 2025,

pose des défis logistiques majeurs, notamment en termes de capacité d’accueil des universités, de qualité de l’encadrement et de disponibilité des terrains de stage. Les facultés doivent s’adapter rapidement pour garantir un niveau de formation élevé malgré l’afflux d’étudiants. Par ailleurs, si l’augmentation du nombre de médecins formés peut, à terme, aider à combler les déficits dans les zones sous dotées, cela dépend également de la mise en place de politiques plus incitatives pour encourager les jeunes médecins à s’installer dans ces régions, voire de la mise en place d’une politique coercitive, comme c’est le cas pour plusieurs professions médicales. Enfin, il nous faut aussi prendre en compte l’impact sociétal : le mode d’exercice de la pratique médicale a largement évolué depuis les années 1970, avec un temps de travail plus faible, comme dans beaucoup d’autres secteurs d’activité. On peut estimer qu’il faut maintenant près de trois jeunes médecins pour remplacer un départ à la retraite. La suppression du est donc un premier pas majeur vers une transformation profonde de la formation médicale en France, même si son effet ne se fera ressentir que dans quelques années.

pour libérer du temps médical, en confiant notamment à des non médecins des activités et des actes aujourd’hui réservés aux médecins. Le précédent gouvernement a beaucoup œuvré en ce sens. Au mois d’avril dernier, l’objectif était de « reconquérir 15 millions à 20 millions de rendez vous chez le médecin » dès 2024. Ces mots ont très vite été suivis d’actions : par décret pris au mois de juin dernier, ce ne sont pas moins de seize procédures qui ont été simplifiées. Ainsi, les pharmaciens peuvent désormais prescrire directement des antibiotiques en cas d’angine ou de cystite. Dans certains cas, il est aussi possible de recevoir une nouvelle ordonnance pour des lunettes directement chez l’opticien. ailleurs, depuis le mois de juin, une expérimentation permettant l’accès direct à un kinésithérapeute ou à un médecin spécialiste, sans passer par un médecin traitant, a été lancée dans treize départements.

Toujours dans l’idée de libérer du temps pour les praticiens, le nombre d’assistants médicaux passera de 6 000 à 10 000 à la fin de l’année. Nous saluons aussi la généralisation du service d’accès aux soins (SAS), effective depuis le mois de juin. Elle vise à répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non programmés de la population partout et à toute heure, grâce à une chaîne de soins lisible et coordonnée entre les acteurs de santé de l’hôpital et de la ville d’un même territoire. Continuer de former davantage de médecins et de soignants, aller chercher des talents à l’étranger et libérer du temps médical : ces trois orientations sont complémentaires. Toutefois, ce débat sur les ressources humaines des professionnels de santé doit s’inscrire dans une stratégie globale, à la fois pour le système de santé et en matière de gestion des ressources humaines. Déterminer le nombre de professionnels à former n’a que peu d’intérêt opérationnel si l’on ne s’assure pas que ceux ci accomplissent effectivement les missions attendues. Par ailleurs, lors d’une audition au mois de mai dernier par la commission des affaires sociales, le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) avait souligné la nécessité d’une évaluation des besoins territoriaux. Madame la ministre, vous l’aurez compris, nous devons travailler ensemble pour coconstruire une feuille de route. Le groupe RDPI

Je donnerai quelques chiffres que vous connaissez certainement sur l’évolution du nombre d’étudiants dans les différentes formations en santé. En médecine, avant 2017, quelque 8 700 places étaient

Pour les professions médicales, le est essentiel afin de redresser la démographie. Mais je vous le dis tout net : le nombre de places ouvertes au concours n’est pas à la hauteur des enjeux. J’ai examiné les projections de très près.

Eh bien, c’est exactement la densité du Limousin en 2012, à une époque où l’on parlait déjà de désertification médicale ! Pour les chirurgiens dentistes, la densité s’accroîtra de 40 % en 2050. Heureuse nouvelle … On atteindra 78 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants. Eh bien, c’est huit de moins que la densité actuelle en région Le plus inquiétant, c’est que ces prévisions ne tiennent pas compte des facteurs sociétaux, de l’évolution des pratiques et de la baisse du temps médical, que l’on a évidemment du mal à évaluer. De surcroît, ces chiffres intègrent le flux des soignants diplômés à l’étranger, sur lequel nous n’avons aucune prise. C’est particulièrement inquiétant pour les chirurgiens dentistes, puisque la moitié, j’y insiste, des inscrits au tableau de l’Ordre cette année sont diplômés de l’étranger. Plutôt

un coup porté à l’excellence universitaire française et une remise en cause de notre souveraineté, puisque, sans ces diplômés étrangers, nous sommes incapables de répondre au besoin de soins de la population. Notre nation aura renoncé à sa capacité de former la totalité des soignants utiles au pays. Il faut donc augmenter le nombre de places au concours, pour atteindre des seuils de densité suffisants bien avant 2050. La massification des étudiants est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante pour résoudre les disparités géographiques. Il faut y associer des dispositifs de régulation : l’État, les pouvoirs publics et le monde universitaire doivent se doter d’une stratégie d’aménagement du territoire – créer des options santé dans les lycées, développer les stages dans les territoires, ouvrir les hôpitaux périphériques aux internes. Bref, il faut se donner les moyens d’une politique déconcentrée pour garantir le déploiement équilibré de l’offre de soins sur le territoire national. Je n’ai malheureusement pas le temps d’aborder la question des pharmaciens, des sages femmes, des kinésithérapeutes, des infirmiers, des aides soignants, autant de professions dont la démographie, le statut ou l’attractivité doivent nous préoccuper. Madame la ministre, former des soignants, c’est investir dans l’humain et dans l’avenir. Le RDSE vous alerte sur la nécessité de recalibrer les ambitions à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer des solutions concrètes. Comment comptez vous vous y pendre ?

2019 a mis en place une planification pluriannuelle du nombre de professionnels à former pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. Des objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour cinq ans – 2021 2025 – ont été ainsi arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après la tenue d’une conférence nationale chargée de présenter des propositions concrètes. Cette première conférence s’est tenue en mars 2021. Il revient ensuite aux universités et aux écoles de maïeutique, en lien avec les agences régionales de santé (ARS), de déterminer le nombre d’étudiants à admettre chaque année

quantitative. Le fixait directement un nombre d’étudiants autorisés à poursuivre dans les études de santé. À l’inverse, la détermination d’objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former implique la concertation des acteurs et impose une approche territoriale d’analyse prospective des besoins en professionnels, en fonction des besoins de santé. Fixer un objectif pluriannuel donne donc plus de latitude aux acteurs locaux. Nous travaillerons en 2025 sur la feuille de

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat proposé aujourd’hui est vaste et difficile à circonscrire. Il ne doit pas nous cantonner dans les idées reçues. Tous ici, dans nos familles, dans nos lieux de vie et dans nos fonctions d’élus, nous constatons la difficulté à accéder aux soins. La question du nombre de soignants formés s’impose. Dans cette situation de pénurie, il serait cependant dangereux d’amalgamer différentes réalités celles des territoires ruraux, où l’accès s’entend aussi au sens littéral du transport vers les lieux de soin, et des zones urbaines ; celles des médecins et des autres soignants ; celles des généralistes et les spécialistes ; celles des soignants de ville et des soignants hospitaliers ; celles des soins urgents et des soins programmés ; celles du secteur public et du système privé. Une évidence s’impose pourtant : l’offre de soins n’est globalement pas à la hauteur de la demande de soins. L’équation n’est pas équilibrée. Alors que l’on raisonne souvent en nombre de soignants formés, je préfère m’en tenir à la seule jauge qui ait du sens : celle du temps de soin effectif.

environ moitié moins de temps médical que leurs aînés. Par un calcul simple, on obtient en fait le temps médical de 6 000 médecins d’il y a quarante ans… Dans ce sens, oui, il faut former encore plus de médecins, en proratisant constamment leur nombre par le temps médical fourni à une population vieillissante, dont les besoins augmentent. Évidemment, cette logique a ses limites : prenons le cas des infirmiers que l’on n’a jamais formés en si grand nombre et qui n’ont jamais eu une durée d’exercice aussi courte, usés sans doute prématurément par leurs conditions de travail. Pourtant, un autre moyen de gagner du temps médical est le report de tâches vers d’autres professionnels de santé, qui doivent eux aussi être en nombre suffisant. La réforme des études médicales est une piste, avec l’arrivée tant attendue, dès l’automne 2026, des fameux docteurs juniors en milieu rural. Ces étudiants en quatrième année de médecine générale approfondiront leur formation tout en apportant du temps médical dans des zones sous dotées. condition de réussite de ce dispositif est cependant la qualité de leur accueil et de leur encadrement, comme le soulignait Corinne Imbert. Pouvez vous me confirmer, madame la ministre, que tout sera prêt en temps et en heure pour accueillir dans les meilleures conditions ces jeunes praticiens ? Une autre piste est celle du temps médical produit par des étudiants français qui font leur cursus à l’étranger. Des passerelles sont elles à l’étude, par exemple pour les jeunes qui sont en Roumanie ou en Espagne, leur permettant de revenir dès les troisième, Peut on leur redonner une possibilité de réussite aux épreuves classantes nationales, qui leur sont quasiment inaccessibles depuis la dernière réforme ? Pour ceux qui sont au delà de la sixième année, donc les internes, favoriser leur retour en France, par exemple en contrepartie d’un exercice en zone sous dense ? Ce serait particulièrement intéressant en cette année qui connaîtra un déficit d’internes… J’évoque enfin, madame la ministre, le cas des médecins en situation de cumul emploi retraite, à qui une exonération totale des cotisations sociales avait été promise. Certains d’entre eux seraient prêts à donner plus de temps médical. Pouvez vous nous confirmer que cette disposition sera prochainement effective dans les termes initialement prévus ? Pour conclure, une chose est certaine : les exonérations fiscales ne donnent pas de temps médical supplémentaire. En revanche, le temps médical des docteurs juniors, le temps médical des docteurs seniors, le temps médical des futurs docteurs, qu’ils soient formés en France ou à l’étranger, le temps de soin en général, toutes professions confondues, sont autant de leviers qui doivent être actionnés simultanément, afin que plus aucun patient, en France, ne se sente abandonné. La

et comment faire en sorte que de jeunes médecins en fin de formation puissent être utiles dans tous les territoires, particulièrement ceux qui sont en difficulté ? Jusqu’à maintenant, la médecine générale était la seule spécialité à n’avoir que trois années d’internat. Cette absence de phase de consolidation était considérée comme une faiblesse, qui ne favorisait pas une installation immédiate en sortie de cursus.

un soutien aux territoires en déprise. Vous avez évoqué des étudiants français qui font leurs études dans des pays européens. Il existe des équivalences qui permettent à ces étudiants de postuler au sein des universités françaises. derniers peuvent également accéder au troisième cycle des études médicales pour effectuer leur formation de spécialité en France. Il leur est

et les années à venir seront encore plus problématiques compte tenu de la vague de départs à la retraite qui nous attend d’ici à 2030. Nous payons aujourd’hui les effets de la politique de non formation d’il y a quarante Il y a donc urgence à former dès à présent beaucoup plus de professionnels de santé et de professionnels paramédicaux, y compris pour faire face au vieillissement de la société et à l’explosion des maladies chroniques. Le remplacement du par le a certes permis d’augmenter le nombre d’internes en médecine, mais cela reste bien insuffisant. Empêcher la démission des personnels passe par une revalorisation des carrières et des rémunérations par l’amélioration des conditions de travail. Dans le même temps, le dogme de la réduction des dépenses publiques appliquée à la santé a fait fuir des dizaines de milliers de soignants, écœurés, lessivés. le cœur de la solution réside dans le budget que vous allez décider d’octroyer aux universités et à notre système de santé tout entier. Ce sera possible si vous résistez aux injonctions de Bruxelles de réduire encore les dépenses publiques, alors que l’Ondam est en hausse quand les besoins nécessiteraient une augmentation de 5 %. Madame la ministre, allez vous expliquer à vos homologues de Bercy que les politiques d’austérité menées pendant des années à l’hôpital sont en grande partie responsables du montant de la facture de la gestion de la covid 19, imputée au budget de la sécurité sociale alors qu’elle aurait dû être supportée par l’État par l’État ? Les services publics et la sécurité sociale doivent être sanctuarisés, au dessus des logiques de réduction de moyens. Or les gouvernements d’Emmanuel Macron ont supprimé 21 000 lits d’hospitalisation, soit 5 % des capacités d’accueil de notre pays.

pour les médecins nouvellement diplômés dans les zones sous denses ». Pour notre part, nous y sommes favorables, tout comme à la régulation des lieux d’installation des médecins et à la réquisition automatique des médecins spécialistes des cliniques privées pour maintenir la permanence des soins.

HD4 vient de cesser ses activités, privant les habitants du département d’une solution qui, si elle était loin d’être idéale, avait le mérite d’exister. Ce n’est pourtant pas faute d’argent public, puisque l’entreprise a empoché 100 000 euros par machine et près de 1,5 million de Les élus sont mis devant le fait accompli et ont dépensé ces sommes pour rien. Mes questions sont donc les suivantes, madame la ministre : allez vous défendre la piste d’une régulation de l’installation ? Allez vous imposer une obligation de participation à la permanence des soins les soirs et les week ends aux professionnels de santé, quel que soit leur mode d’exercice ? Allez vous défendre l’idée

! Compte tenu des voies de contournement existantes – départ pour un pays étranger, choix d’une autre activité professionnelle, déconventionnement… –, le risque est important de voir cette pénurie s’aggraver encore. Je rappelle que le PLFSS pour 2022 a permis à chaque profession d’inclure des mesures de régulation démographiques dans ses négociations conventionnelles

madame la ministre, mes chers collègues, alors que nous débattons, près de 8 000 étudiants en médecine révisent les épreuves dématérialisées nationales (EDN) qui commenceront dans six jours. À l’issue du concours, 7 974 étudiants se verront attribuer une place en internat dans les différentes spécialités, ce qui représente 1 510 postes d’internes en médecine de moins que l’an dernier. Et pour cause,

et étudiantes. C’est sur cette faible somme que reposait la promesse illusoire de voir s’ouvrir de nouvelles places en deuxième année de médecine. Madame la ministre, l’ARS et les facultés de médecine, désormais chargées d’arrêter les objectifs pluriannuels d’admission, sont à court de moyens pour augmenter les places, alors que les facultés sont déjà largement saturées. Et pour cause, l’augmentation du nombre d’étudiants, d’étudiants, qui constitue déjà un enjeu en soi, doit s’articuler avec une capacité d’accueil dans les lieux de stage – vous l’avez dit tout à l’heure. Ainsi, en 2024, soit quatre ans après la réforme, nous avons seulement

les 6 000 généralistes demandés par les maires ruraux ni de pourvoir les 30 % de postes de psychiatres hospitaliers vacants ! Cela fera encore moins revenir les 700 médecins généralistes qui sont partis à la retraite en 2023

plus précisément et avec transparence. Par ailleurs, le financement de la réforme d’entrée dans les études de santé (Rees) devra s’accompagner de réformes similaires pour l’intégralité des professions soignantes : infirmiers, aides soignants, sages femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes… En effet, la réalité est que nous manquons de toutes ces professions. Et parce qu’augmenter les places en formation ne suffira pas à attirer plus d’étudiants en formation, il faudra créer des écoles normales des métiers de

à exercer dans les territoires sous dotés en offre de soins. Les écoles normales des métiers de la santé représentent un double investissement, pour l’accès aux soins et pour les étudiants en santé. d’abord, ces écoles permettraient d’accroître le nombre de soignants, d’éradiquer les déserts médicaux et de garantir l’accès aux soins. Ensuite, elles permettraient aux étudiants de poursuivre des études de santé sans condition de ressources, de garantir l’égalité des chances et la diversité socio économique et de revaloriser des professions délaissées. Pour rappel, une formation d’aide soignant coûte entre 6 000 euros et 10 000 euros à l’étudiant lui même, pour un salaire inférieur à 2 000 euros en début de carrière. Comment penser attirer des professionnels du quand ils doivent payer aussi cher pour se former ? Nous le devons à celles et ceux qui travaillent tous les jours pour notre santé et pour celle de nos proches : investissons dans la formation des professionnels de santé et dans l’accès aux soins !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord moi aussi à remercier nos collègues du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky d’avoir inscrit ce débat fondamental à l’ordre du jour de notre assemblée.

de longue durée (ALD) n’ont pas de médecin traitant, ce qui est particulièrement grave. C’est donc la promesse d’égalité d’accès à la santé, au cœur de notre modèle social, qui est brisée pour de nombreux Français. Confrontés chaque jour au désarroi de nos

qui ont pris des arrêtés mettant en demeure l’État de lancer dans les plus brefs délais un plan d’urgence pour l’accès à la santé, invoquant le respect de la dignité de la personne humaine. Ce constat de la pénurie est établi et documenté depuis de nombreuses années. Pour autant, le manque de soignants – médecins, infirmiers, sages femmes, aides soignants – ne cesse de progresser et aboutit à des situations souvent dramatiques. En témoigne l’état dans lequel se sont encore trouvées les urgences cet été dans notre pays.

Le Premier ministre a annoncé que la santé mentale serait l’une des causes de l’année, mais avec quels moyens, madame la ministre ? Cela semble extrêmement compliqué… Si l’augmentation des effectifs en formation est une nécessité, elle doit absolument tenir compte des effectifs d’étudiants qui pratiquent réellement la médecine en fin de cursus, de l’évolution des pratiques médicales, de l’évolution démographique de la société, des besoins réels des territoires et et des spécialités sous dotées. Et il faut, bien sûr, une politique budgétaire qui aille en ce sens ! L’ambition affichée par le précédent gouvernement est de passer à 12 000, puis à 16 000 élèves, mais, vous l’avez dit, il ne suffit pas de décréter un chiffre – ce serait trop simple. Il faut aussi donner les moyens. Lesquels ?

de former davantage de soignants a un corollaire : celui d’augmenter les moyens des universités. Au reste, il n’y a pas que le nombre : comme l’ont souligné plusieurs de mes collègues, il faut augmenter et diversifier les lieux de stage de médecine, notamment dans les zones sous denses, et former plus de maîtres de stage universitaire,

un médecin a deux fois plus de chances de s’installer dans une zone sous dotée s’il en est originaire ou s’il y a été scolarisé. Il faut également généraliser l’initiative intéressante de la région Occitanie, qui a créé dès le lycée une spécialité santé, pour susciter des vocations pour tous les métiers de la santé, au delà de la seule médecine.

Outre les médecins, la France connaît une pénurie d’infirmiers et d’aides soignants, puisque ces deux professions sont confrontées à une baisse de leur attractivité due aux conditions de travail de plus en plus difficiles : manque de personnel, manque de reconnaissance, horaires décalés, etc. Là encore, la sonnette d’alarme a été tirée depuis longtemps, mais, si le Ségur de la santé est venu revaloriser financièrement ces professions, rien n’a été fait pour améliorer ces conditions de travail. Ainsi, près de 200 000 infirmiers diplômés n’exercent plus,

Selon cette étude et au regard des besoins de notre population, le nombre de jeunes diplômés couvrirait moins des deux tiers des besoins en aides soignants. Nous le voyons, mes chers collègues, il est plus que nécessaire de former plus de soignants.

créer une organisation territoriale qui mette fin aux inégalités majeures et insupportables existant aujourd’hui. Face à cette situation, que les Français vivent comme un véritable déclassement, nous attendons des réponses rapides. Il ne suffira pas d’appeler à la rescousse les médecins retraités, qui sont déjà aujourd’hui

J’y souscris pleinement, mais cela ne doit pas éluder un défi tout aussi essentiel : comment faire en sorte que ces médecins s’installent dans les territoires qui en ont le plus besoin ? Comment utiliser leur formation comme un levier de résorption des inégalités territoriales d’accès aux soins ? j’ai entendu nombre de parties prenantes et de professionnels, en tant que rapporteur de la mission d’information sur les inégalités territoriales d’accès aux soins dans le cadre de la commission de l’aménagement du territoire et Les enseignements que j’en retire permettent d’esquisser pour l’avenir des pistes que j’aimerais partager avec vous. Une première réponse réside dans l’évolution de la sélection, pour favoriser le recrutement en médecine d’étudiants issus de zones sous dotées. La ruralité et les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont largement sous représentés parmi les territoires dont sont issus les étudiants en santé. Or ceux ci sont les plus enclins à s’installer dans ces espaces à l’offre de soins insuffisante. Pourquoi ne pas définir des taux minimaux d’étudiants issus de ces territoires, comme c’est déjà le cas pour les boursiers ? Un tel dispositif serait plus efficace que le très cher contrat d’engagement de service public, aux résultats aujourd’hui insuffisants. Il faut en outre mener un véritable choc de territorialisation de la formation. Les futurs professionnels de santé s’ancrent progressivement dans leur territoire de formation lors de leurs études et s’installent souvent à proximité.

Ce virage territorial doit également s’appliquer aux stages, pour sortir de notre modèle trop « CHU centré ». Davantage de stages doivent être réalisés en médecine de ville, pour permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux lieux d’exercice et méthodes de travail, en particulier dans les maisons de santé. Faire venir les jeunes dans les territoires sous dotés est une clé pour répondre aux disparités territoriales. Bien sûr, un tel changement de logiciel suppose de mieux accompagner nos étudiants, notamment en mettant en place des indemnités de déplacement et de logement suffisantes. Enfin, il faut lever le tabou de la régulation des installations. La situation actuelle est le résultat de décennies d’incitations financières des médecins à s’installer en zone sous dense. Le bilan est sans appel un accroissement des inégalités d’accès aux soins et 6 millions de Français sans médecin traitant. Cessons enfin de distribuer vainement l’argent public ! Une régulation pourrait être instaurée pour les étudiants à l’issue de leur formation, en ouvrant la possibilité d’installation en zone mieux dotée seulement lors du départ d’un médecin, ou

je vous remercie

Les temps d’attente atteignent plusieurs semaines, au minimum, pour un généraliste, et plusieurs mois pour un spécialiste. Ce phénomène n’est, bien entendu, pas homogène : certains territoires s’en sortent mieux, alors que d’autres sont devenus de véritables déserts médicaux. Le législateur a bien pris conscience de l’ampleur de cette crise en supprimant, en 2019, le qui limitait le nombre d’étudiants en médecine.

C’est pourquoi, dans l’immédiat, nous devons faire preuve d’imagination et de pragmatisme pour apporter des solutions à la pénurie de médecins et de soignants. À court terme, le Gouvernement a fait le choix de déléguer de plus en plus de tâches médicales aux infirmiers, aux aides soignants et à d’autres professionnels de santé. Ces délégations d’actes comprennent, par exemple, la prescription et l’administration de vaccins par les infirmiers, ou encore le renouvellement, par les pharmaciens, d’ordonnances pour les maladies chroniques. Ouvrir plus largement les délégations d’actes était sans doute une mesure nécessaire pour permettre à notre système de santé de faire face à la demande de soins. Mais prenons garde : on peut déléguer à condition que cela ne morde pas sur le temps médical accordé aux patients.

Il ne faudrait pas priver le patient du temps médical dont il a besoin. Par ailleurs, les infirmiers et les aides soignants sont, eux mêmes, en sous effectif. Ils sont épuisés. Leurs horaires et leur charge de travail s’alourdissent considérablement, cela pourrait, à terme, nuire à la qualité des soins qu’ils prodiguent. On ne peut donc pas continuer à leur déléguer toujours plus d’actes. Ainsi, madame la ministre, cette réponse de court terme ne peut être satisfaisante. Elle a ses limites, et nous ne pouvons continuer à faire peser tout le poids de la crise sur les épaules de nos soignants. Si cette solution permet de tenir dans l’immédiat, il est nécessaire de trouver d’autres pistes. Surtout, il nous faut penser au long terme. Il est impératif de remédier, de manière structurelle, au manque d’offre de soins dans notre pays, en formant plus de médecins. Mais cela pose plusieurs problèmes, auxquels la fin du ne répond pas complètement. Il y a d’abord la question des places disponibles dans nos universités de médecine. Nos facultés ne peuvent accueillir un nombre d’étudiants infini. Le a d’ailleurs notamment pour but de s’assurer que le nombre d’étudiants admis est cohérent avec la capacité d’accueil de chaque faculté. Pour former plus d’étudiants, il faudrait plus de moyens. Or la situation de nos finances publiques ne semble pas nous le permettre. Ensuite, un problème de ressources humaines se pose. La médecine est un art qui se transmet. Pour former de nouveaux médecins, encore faut il avoir des professeurs pour enseigner aux étudiants, et des médecins expérimentés pour encadrer les internes. Or, sous l’effet des départs à la retraite, le nombre de praticiens expérimentés diminue, et ceux qui restent sont désormais surchargés. Comment, dans ces conditions, réussir à former en nombre suffisant une nouvelle génération de médecins compétents ? Madame la ministre, le gouvernement auquel vous appartenez aura donc une double responsabilité. d’abord, à long terme, il devra trouver les moyens humains et financiers pour former une nouvelle génération de médecins et de soignants. Ensuite, à court terme, il lui faudra trouver des solutions innovantes pour répondre au manque au manque de médecins et de soignants sur notre territoire, car nos citoyens ont besoin d’accéder à ces soins sans attendre. La parole est à Mme

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la formation des soignants constitue malheureusement une préoccupation phare de notre société. Cette problématique s’étend et inquiète bien au delà du domaine médical et paramédical. Abandon de cursus, problèmes de recrutement, départs vers le privé : ces maux, dont souffre l’ensemble du corps médical, sont bien connus. Ils constituent une affection de longue durée, qui perdure d’année en année au sein de notre société. Pour autant, nous avons récemment pu entrevoir les prémices d’une rémission en la matière. D’après les chiffres publiés par le Conseil national de l’ordre des médecins au début du mois d’octobre, 1 672 médecins supplémentaires sont entrés en fonction au cours de l’année 2024, soit une hausse de 0,8 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, malgré cette éclaircie, les déserts médicaux, dans nos villes et dans nos campagnes, eux, progressent. Dans le département dont je suis élue, l’Ardèche, 35 000 personnes n’ont pas accès à un médecin traitant. Ce constat n’est pas nouveau. Il est la conjugaison de plusieurs facteurs, certains maîtrisables, d’autres inéluctables. Parmi les écueils à l’origine de la catastrophe quotidienne que vivent tant de nos concitoyens, deux, en particulier, doivent être rappelés. Notre première erreur a été de former toujours moins de médecins chaque année. Le, dont la suppression a été trop tardive, a durablement affecté le renouvellement générationnel, particulièrement celui de nos soignants de proximité.

D’ici là, les zones déjà sous dotées continueront inexorablement de voir les départs de leurs médecins non compensés et leur population privée d’un accès aux soins minimum. Notre seconde erreur a été le choix d’une organisation centrée sur l’hôpital, qui concentre l’activité des soins et qui contribue ainsi à accroître une répartition déjà inégale de l’offre sur le territoire. Face à ce fléau qui gangrène nos communes et leur fait perdre petit à petit leur attractivité, nos élus locaux ont été fidèles à l’ingéniosité et au sens pratique qui les caractérisent tant. Je pense notamment à la création de maisons de santé pluridisciplinaires et au recrutement de personnels déchargeant les médecins des tâches administratives. Malheureusement, les initiatives concrètes et innovantes pour lutter contre les les déserts médicaux, souvent engagées avec détermination par les collectivités locales, mais isolées, ne peuvent à elles seules résoudre cette problématique. Sur ce sujet comme sur tant d’autres, écouter les propositions de la Haute Assemblée aurait permis un gain de temps non négligeable. En effet, le 18 octobre 2022, le Sénat adoptait la proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine Présenté par notre ancien président Bruno Retailleau, que je tiens à saluer, ce texte cherchait à agir au moment de la formation des médecins en créant une quatrième année d’internat. L’objectif était ainsi d’inciter les jeunes médecins à effectuer leur dernière année de formation dans des zones sous dotées en cabinet libéral ou en maison de santé, avec une rémunération à l’acte. ait été dénaturé, le dispositif a été retenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, et la première promotion concernée a fait sa rentrée en 2023. Madame la ministre, quels sont les premiers enseignements que nous pouvons tirer de ce dispositif ? ? Comment allez vous assurer le déploiement effectif et rapide des assistants médicaux, des 2 000 nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires et des bus de santé, promis par le Premier ministre ? La parole

Cette tension est la conséquence à la fois d’une évolution des besoins de santé, supérieurs aux capacités de formation, d’un nouveau rapport au travail et aux conditions de son exercice, mais aussi d’une répartition insuffisamment efficace des professionnels entre les différents offreurs de soins. De manière prospective, la poursuite du vieillissement de la population et l’absence de perspective de diminution du nombre de personnes touchées par les grandes causes de morbidité laissent présager un besoin croissant de professionnels de santé.

qui permet d’analyser la situation du point de vue des ressources humaines pour la totalité de l’année 2023. Celle ci révèle plusieurs signaux positifs sur le plan de l’attractivité des métiers hospitaliers, ce qui confirme que l’attention portée à la rémunération, mais aussi aux conditions de travail, porte ses fruits.

L’absentéisme continue également de décroître, pour s’établir, tous établissements confondus, à 9,5 %, contre 11,1 % en 2022, soit le niveau le plus bas observé depuis la covid Dans cette situation, bien sûr, la priorité doit être de soutenir la reconquête progressive de l’attractivité des métiers de la santé et de la fidélisation des professionnels. Les études en santé – médecine, pharmacie et formation en soins infirmiers – occupent le podium des formations les plus demandées par les lycéens sur Parcoursup en 2024. Il faut le souligner, ce sont des métiers qui attirent. Afin de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, le Gouvernement a engagé des mesures fortes ces cinq dernières années pour accroître ses capacités de formation, mais aussi maintenir dans le système de santé les étudiants formés et les professionnels en exercice.

Cette transformation implique l’accès direct à de nouvelles professions de santé, mobilisant notamment les nouveaux métiers paramédicaux, ainsi que l’élargissement des compétences des professionnels de santé. Les protocoles de coopération, locaux et nationaux, bien qu’ils soient

clairement en faveur d’un très grand effort de formation. Je souligne, car, il y a encore quelque temps, sûrement en toute bonne foi,

Merci